La séance est ouverte. Le compte rendu intégral de la séance du mercredi 18 décembre 2019 a été publié sur le site internet du Sénat. Il n'y a pas d'observation ? ... Le procès-verbal est adopté. j'ai le regret de vous faire part du décès de notre ancien collègue François Autain, qui fut sénateur de la Loire-Atlantique de 1983 à 2011. demande du groupe Les Républicains, sur l'avenir des transports express régionaux. Nous allons procéder au débat sous la forme d'une série de questions-réponses dont les modalités ont été fixées par la conférence des présidents.

Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, les transports express régionaux (TER) sont un élément essentiel du maillage de nos territoires. En France, 7 000 trains TER circulent sur 20 000 kilomètres de lignes de chemin de fer, dont 9 000 kilomètres de lignes de desserte fine du territoire, sans oublier les 1 300 autocars qui complètent cette offre de mobilité. Ils transportent chaque jour quelque 900 000 voyageurs. Grâce aux financements des autorités organisatrices régionales, l'offre TER a progressé de plus de 25 % depuis 1997, et le trafic a crû de plus de 50 %. Malgré ce rôle essentiel de maillage, notamment dans les territoires ruraux, où l'offre de mobilité est réduite, les TER souffrent aujourd'hui de nombreux maux, qui nous amènent à nous interroger sur leur pérennité. En effet, ils subissent une baisse de fréquentation qui s'explique essentiellement par le manque de régularité du réseau : des trains en retard ou supprimés, ou encore des incidents d'exploitation. Alors que nous évoquons l'intermodalité dans les transports et la nécessité de faire du transport ferroviaire la colonne vertébrale de cette dernière, une telle tendance ne peut que nous alarmer. Ce manque de régularité a une cause très claire, soulignée d'ailleurs par le récent rapport de la Cour des comptes : il s'agit de l'état très dégradé du réseau. En janvier 2019, SNCF Réseau indiquait que seuls 29 % de ces lignes régionales étaient jugées en bon état, tandis que plus de la moitié était touchée par des ralentissements, voire par une suspension de service. Un rapport sur les lignes de desserte fine du préfet François Philizot est d'ailleurs très attendu par l'ensemble des élus et des acteurs de la mobilité. Dans le cadre de la rédaction du rapport sur la loi du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités (LOM), j'avais pu auditionner le préfet Philizot. Selon lui, 7,4 milliards d'euros seraient nécessaires pour remettre en état l'ensemble de nos petites lignes ferroviaires. C'est une somme colossale, qui nous amène à nous interroger sur le manque de moyens consacré dans le temps à l'entretien de notre réseau ferré. Si un tel coût venait à se confirmer, le budget de l'Agence de financement des Les TER sont aujourd'hui majoritairement couverts par la subvention des régions, à hauteur de 3,1 milliards d'euros, et par les voyageurs, à hauteur de 1 milliard d'euros. La Cour des comptes pointe, là aussi, une hausse continue des coûts d'exploitation depuis 2012. Ainsi, les coûts complets d'exploitation, en comptant l'impact environnemental et le régime de retraite des cheminots- sujet d'actualité -, s'élevaient à 8,5 milliards d'euros en 2017, dont le financement était assuré à 88 % par des subventions publiques. L'État avait d'ailleurs indiqué son souhait de se désengager des petites lignes en demandant à SNCF Réseau, dans son contrat de performance, de ne plus investir sur ce segment et en réduisant son intervention dans le cadre des contrats de plan État-région Logiquement, les régions sont désormais seules en première ligne pour maintenir cette offre de mobilité dans les territoires, et ce dans le cadre de budgets de plus en plus restreints. Néanmoins, des réformes majeures engagées ces dernières années devraient aider les régions à améliorer cette offre de mobilité et permettre au TER de regagner en attractivité. 2018 pour un nouveau pacte ferroviaire prévoit l'ouverture à la concurrence des services non conventionnés à partir du 1 janvier 2019, en vue d'une exploitation à partir de décembre 2020. à partir de décembre 2020. Depuis le 3 décembre 2019, et jusqu'au 23 décembre 2023, l'État et les régions pourront ainsi attribuer des contrats de service public de transport ferroviaire de personnes, après publicité et mise en concurrence.

Le Sénat a joué un rôle clé dans la préparation de cette réforme, avec l'adoption en mars 2018 de la proposition de loi d'Hervé Maurey et de Louis Nègre relative à l'ouverture à la concurrence du transport ferroviaire de voyageurs. Grâce à cette proposition de loi, nous avons pu coconstruire, en bonne intelligence avec le Gouvernement, le projet de loi pour un nouveau pacte ferroviaire. Enfin, lors de l'examen de la loi d'orientation des mobilités, le Sénat a réaffirmé son engagement pour les lignes à desserte fine, qui représentent une offre de mobilité indispensable. La LOM répond d'ailleurs à une des préconisations de la Cour des comptes et clarifie les rôles entre l'État, les régions et le gestionnaire d'infrastructure. Ainsi, concernant les lignes de desserte fine, la LOM prévoit la possibilité de transférer leur gestion aux régions qui en feraient la demande.

Bien entendu, ce transfert de compétence ne règle pas le problème du manque d'investissement de l'État, afin d'accompagner les régions dans cette offre de mobilité. De même, l'ouverture à la concurrence ne pourra pas apporter une solution miracle à tous ces problèmes, notamment le coût de régénération du réseau ferré. Ainsi, nombre de ces lignes de desserte fine sont aujourd'hui menacées, et il appartiendra aux régions d'évaluer la pertinence de conserver chacune d'entre elles, selon les spécificités de chaque territoire. de son rôle auprès des collectivités territoriales, continuera de veiller à l'avenir de ces petites lignes, qui permettent à nos territoires ruraux de sortir des zones blanches de la mobilité et à nos concitoyens de bénéficier d'une offre de mobilité

Monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, avec cette nouvelle année, pour laquelle je vous présente mes meilleurs voeux, entrent en vigueur plusieurs dispositions majeures issues du nouveau pacte ferroviaire voté en 2018, dans le plus strict respect des engagements pris par le Gouvernement. la SNCF est depuis le 1 janvier un groupe public unifié, constitué de sociétés nationales à capitaux publics. En recréant un groupe plus intégré, il s'agit d'améliorer l'efficacité opérationnelle de la SNCF, pour en faire une entreprise apte à affronter les enjeux de demain. La loi de finances pour 2020, qui vient d'être adoptée, organise la reprise de 25 milliards d'euros de dettes de SNCF Réseau. C'est un effort sans précédent pour notre système ferroviaire, qui doit permettre à ce dernier de retrouver une trajectoire soutenable : dès cette année, plus de 400 millions d'euros de frais financiers seront économisés et réinjectés dans la rénovation du réseau ; ce point me paraît essentiel à souligner. La fin du recrutement au statut de cheminot est par ailleurs effective depuis le 1 janvier dernier. Enfin, et cela fait cela fait directement le lien avec notre débat d'aujourd'hui, l'État et les régions sont depuis le 3 décembre libres de mettre en concurrence l'exploitation des services qu'ils organisent, respectivement les trains Le train express régional transporte chaque jour près de 1,3 million de voyageurs dans environ 7 900 trains et 1 300 autocars. Il s'agit donc d'un maillon essentiel des transports du quotidien pour nos concitoyens, sur l'ensemble du territoire national, comme cela a été rappelé par M. Mandelli. Je tiens à rappeler que les TER sont et resteront des services conventionnés, c'est-à-dire déficitaires et subventionnés par de l'argent public. C'est vrai pour absolument toutes les lignes, avec un taux de subvention du contribuable de 75 % en moyenne à l'échelle nationale, les recettes des billets couvrant les 25 % restants, moins que dans la plupart des pays européens. En 2019, les régions ont versé environ 3 milliards d'euros de subventions d'exploitation à la SNCF. Avec l'ouverture à la concurrence, ce principe ne changera pas il ne s'agit nullement d'une privatisation, comme on a pu l'entendre dire à tort ici et là. Les régions resteront aux commandes de ces services publics, dont elles continueront de définir l'ensemble des aspects : dessertes, horaires, confort, tarifs, services à bord et en gare. Ainsi, il ne revient pas à l'État de se substituer aux régions, à qui appartient le suivi de la performance des services qu'elles organisent, en vertu du principe constitutionnel de libre administration des collectivités territoriales, auquel je sais votre assemblée spécialement attachée. Par ailleurs, l'amélioration de la productivité constitue un enjeu fondamental pour la compétitivité du transport ferroviaire par rapport aux autres modes de transport et une préoccupation majeure d'acteurs tels que la Cour des comptes, préoccupation sur laquelle je reviendrai plus tard. Cet objectif relève avant tout du management de SNCF Voyages, entreprise publique. En particulier, la négociation des conditions de travail participe des prérogatives des partenaires sociaux, et il ne revient pas à l'État de remettre en cause ce que ceux-ci négocient, dans le respect du cadre posé par le pacte ferroviaire. Le rôle de l'État est de créer les conditions optimales pour favoriser l'attractivité du mode ferroviaire. C'est bien ce qui guide l'action du Gouvernement depuis 2017. Ainsi, l'ouverture du secteur ferroviaire à la concurrence permettra d'offrir aux voyageurs de nouveaux services, au meilleur coût. L'État travaille à préparer le système ferroviaire à cette ouverture en fixant les règles pour que celle-ci puisse s'exprimer dans des conditions équitables entre tous les opérateurs. De nombreux textes d'application ont ainsi été publiés au cours des dix-huit derniers mois, après concertation avec l'ensemble des acteurs. En ce qui concerne l'organisation de la SNCF, le choix de faire de SNCF Voyages une société à part entière lui offrira la flexibilité nécessaire pour adapter son organisation en fonction de ses besoins. En particulier, l'entreprise aura désormais le choix d'exploiter ses services nationaux directement ou à travers des filiales. Sur le plan social, l'État a engagé la création d'un nouveau cadre harmonisé pour les salariés du transport ferroviaire. Au-delà de la fin des embauches au statut, cela se traduit par les négociations en cours entre les partenaires sociaux sur la convention collective de branche, que le Gouvernement veut de haut niveau. Enfin, en ce qui concerne les infrastructures, comme je l'ai souligné en introduction, l'État a consenti un effort sans précédent avec la reprise de 35 milliards d'euros de dette de SNCF Réseau, 25 milliards d'euros au 1 janvier 2020. À terme, cela permettra à SNCF Réseau d'économiser de l'ordre de 1 milliard d'euros par an de frais financiers, donc d'intensifier ses investissements en faveur de la remise en état de ses infrastructures ferroviaires sans dégrader sa situation financière. Je vous rappelle que 3,6 milliards d'euros par an sur dix ans, auxquels s'ajouteront 200 millions d'euros par an à partir de 2022, seront ainsi consacrés aux investissements de régénération du réseau ferré national, qui représentent aujourd'hui 90 % des circulations et 80 % des circulations de TER. Cela correspond à une hausse de 50 % par rapport à la précédente de 50 % par rapport à la précédente décennie. S'agissant des petites lignes ferroviaires, dont les investissements de régénération sont pris en charge par l'État et les collectivités dans le cadre des il convient de rappeler que leur coût complet, en incluant les dépenses d'entretien et d'exploitation, reste financé aujourd'hui par l'État et par SNCF Réseau à plus de 70 %, en tenant compte de l'effort accru des régions ces dernières années pour cofinancer les investissements nécessaires à leur remise en état. Nous sommes tous conscients ici de la nécessité de faire face à un pic d'investissements historique pour la décennie à venir sur ces lignes, dont les rails et les plateformes sont arrivés au terme de leur durée de vie. au terme de leur durée de vie. Cela représente plusieurs centaines de millions d'euros par an au cours des prochaines années, pour lesquels je tiens à vous confirmer, d'une part, que le Gouvernement respectera les engagements pris par l'État dans le cadre des CPER actuels, prolongés jusqu'à la et, d'autre part, que les travaux du préfet Philizot, menés en partenariat avec les régions, ont permis de recenser l'ensemble des besoins et de bâtir des plans d'action régionaux, qui seront signés dans les prochaines semaines, avec des solutions innovantes et adaptées à chaque ligne, en termes techniques et de gouvernance. Ces solutions pourront notamment s'appuyer sur les possibilités introduites par l'article 172 de la LOM, qui ouvre par exemple la voie à des transferts de gestion de certaines petites lignes au profit des régions qui en feraient la demande. En parallèle, je souhaite que l'État impulse la création d'une véritable filière de « trains légers », pour redonner au TER la place qu'il mérite, y compris sur des dessertes fines des territoires. En jouant simultanément sur le dimensionnement des infrastructures, de la signalisation et des matériels roulants, je suis convaincu que des économies de l'ordre de 30 % à 40 % sont réalisables, en investissement comme en exploitation. Ces nouvelles possibilités permettront de mieux faire face aux besoins de chaque territoire, en fonction du contexte et des besoins identifiés par les acteurs locaux en matière de transport public. En cela, le Gouvernement répond pleinement à la première recommandation du rapport que la Cour des comptes a rendu public à l'automne 2019 sur la gestion des TER entre 2012 et 2017. Pour terminer, je souhaite revenir quelques instants sur ce rapport, qui a pu faire l'objet d'interprétations caricaturales, à commencer par le niveau d'engagement de l'État en faveur du ferroviaire. Des neuf recommandations de la Cour, seules deux impliquent directement l'État : la première, que j'évoquais à l'instant, et la septième, relative à la disponibilité des données afin de réussir l'ouverture à la concurrence. Cette seconde recommandation a été également satisfaite, à travers le décret Données, publié cet été pour permettre à l'État, pour les TET, et aux régions volontaires de préparer les premiers appels d'offres : il s'agit des régions Grand Est, Provence-Alpes-Côte d'Azur et Hauts-de-France. Toutes les autres recommandations de la Cour s'adressent aux régions et à la SNCF. Elles concernent notamment la qualité du service, les analyses socioéconomiques, les coûts d'exploitation, le niveau de présence des agents en niveau de présence des agents en gare et à bord, les plans de transport, la tarification, l'expertise des régions ou encore l'organisation interne de l'activité TER à la SNCF. Il faut

Je rappelle que chaque orateur dispose de deux minutes au maximum pour présenter sa question, suivie d'une réponse du Gouvernement pour une durée équivalente. Dans le cas où l'auteur de la question souhaite répliquer, il dispose de trente secondes supplémentaires, à la condition que le temps initial de deux minutes n'ait pas été dépassé.

l'entreprise. SNCF Réseau n'est pas dans la trajectoire prévue. Bien sûr, et je l'avais souligné, la dette a été reprise. Félicitations ! Mais, si je m'en tiens à l'avis qu'elle a rendu le 19 décembre, l'Autorité de régulation des transports s'inquiète fortement du non-respect de la trajectoire financière le contrat de performance SNCF Réseau 2017-2026 et de l'insuffisance des investissements de renouvellement du réseau,

Monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, en Auvergne, les lignes d'irrigation du territoire représentent 60 % du réseau ferroviaire. C'est dire l'importance qu'elles revêtent pour assurer la desserte de territoires fortement enclavés. Or leur coût fait peser le risque d'une fermeture totale ou partielle de certaines d'entre elles. Si une étude approfondie et impartiale de la fréquentation de chaque ligne doit, de toute évidence, être menée, ce seul critère, bien sûr très pénalisant en zone rurale, ne saurait être retenu, d'autant plus que cette appréciation peut se révéler subjective. En effet, le rapport de la Cour des comptes, publié en octobre 2019, portant sur l'avenir des TER souligne une diminution de leur fréquentation sur la période 2012-2018 à l'échelon national : nous pourrions y voir surtout une stagnation après une forte hausse sur la période précédente, due aux efforts des régions ; cela correspond également à une stabilisation de l'offre de transport, qui avait également évolué. En ce qui concerne les explications apportées, à savoir la dégradation continue de la qualité du service pour partie liée à un mauvais état du réseau, nous les partageons. En Auvergne, le réseau est électrifié à Ce sont là, pour nous, les véritables causes de la baisse de fréquentation de ces petites lignes. Aussi, plutôt que d'aborder la question à travers le seul prisme de l'analyse économique, nous espérons que l'utilité sociale et environnementale sera prise en compte pour juger de la pertinence Dans le cadre du plan de sauvegarde des lignes d'irrigation du territoire de la région Auvergne-Rhône-Alpes, adopté en 2016, la contribution de 50 millions d'euros prévue pour l'État est insuffisante. Malgré les efforts de la région, qui apporte trois fois plus, sa réalisation est donc incertaine. Monsieur le secrétaire d'État, pourriez-vous rassurer nos concitoyens, en confirmant que l'État soutiendra les petites lignes pour mettre fin au contre-report modal et répondre à leurs besoins en mobilité ?

Bernard Buis. Monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, depuis un mois, les régions peuvent organiser des appels d'offres pour l'exploitation de lignes de trains express régionaux. Cette ouverture progressive à la concurrence des lignes de TER, instituée par le pacte ferroviaire, a été saluée par le rapport thématique de la Cour des comptes, publié en octobre dernier. Celui-ci définit cette évolution comme un facteur essentiel de réussite du TER. La réussite des TER est fondamentale, car elle conditionne le maillage, la vitalité et la cohésion des territoires auxquels ce type de mobilité a vocation à concourir. Ce point est justement au coeur de l'action du Gouvernement, dans les choix qu'il a faits. Rappelons qu'il avait écarté, dans le cadre du pacte ferroviaire, la préconisation du rapport Spinetta relative à la fermeture de lignes peu fréquentées. Je mesure bien ce que veut dire le maintien d'une ligne dans un territoire pour ses étudiants, ses lycéens, ses salariés ou encore ses touristes pour rejoindre des lignes centres. Il me plaît de souligner votre engagement pour la ligne Grenoble-Veynes et l'engagement de l'État lors du tour de table financier pour assurer la régénérescence de cette ligne. Monsieur le secrétaire d'État, je vous en remercie. dans son rapport : une suppression n'est pas la seule solution. Il préconise à ce titre que soit réalisée une analyse sociale, économique et objective des lignes peu fréquentées, pour permettre aux régions de choisir entre plusieurs options sur leur devenir. En effet, En effet, la fréquentation ou la rentabilité ne peut être l'unique critère du maintien ou du non-maintien d'une desserte ferroviaire quand celle-ci est indispensable à la vie d'un territoire. C'est d'ailleurs là la raison même d'être d'un service public. Monsieur le secrétaire d'État, vous avez accueilli plutôt favorablement cette recommandation. Si l'arbitrage sur l'offre des services TER revient à la région, comment le Gouvernement entend-il éclairer, notamment par l'expertise technique des services de l'État, cette prise de décision, afin qu'elle ne freine pas la réduction de la fracture territoriale ? Aussi, dans quelle mesure estimez-vous que l'ouverture à la concurrence généralisée en 2023 dans les TER aura un impact sur le maintien ou non des lignes peu fréquentées ?

ceux que j'ai évoqués dans mon propos liminaire sur la transmission des données, de manière que les entreprises ferroviaires, les régions et l'ensemble des parties prenantes puissent avoir accès aux informations nécessaires afin de concevoir les offres qui, plus tard, feront l'objet d'une convention de service public avec Enfin, je vous remercie de votre mot sur Grenoble-Veynes. C'est effectivement un dossier important, car il s'agit d'une ligne structurante, sur laquelle un premier accord de financement a été conclu. L'État prendra sa part, en lien avec les différents acteurs du territoire, pour pérenniser une ligne qui est à la fois belle et nécessaire.

depuis le mois dernier, les régions peuvent lancer des appels d'offres pour les TER. Vous le savez, nous avons combattu cette disposition du pacte ferroviaire.

Nous ne croyons pas que la libéralisation entraînera une progression de la qualité du service aux usagers. L'ensemble des expériences européennes nous donne d'ailleurs raison, et ce n'est pas pour rien que les Britanniques souhaitent faire marche arrière. Nous considérons que la dimension territoriale nationale de la SNCF est un atout à préserver. Perdre cela, c'est mettre à mal le caractère universel du droit à la mobilité. Nous croyons que la solution est ailleurs, par exemple dans une implication plus grande des régions et des usagers au sein même de la gouvernance de cette société à 100 % publique, cette démocratisation s'appuyant sur des objectifs de présence territoriale renforcée, et non, comme le soutient la Cour des comptes, sur l'abandon de certains tronçons. Par ailleurs, comment penser que changer d'opérateur tout en gardant des réseaux vétustes permettra une quelconque amélioration de l'offre ? Comment croire que, en période de disette budgétaire, les régions ne vont pas chercher à faire des économies en donnant prime au moins-disant social, environnemental et économique, voire en taillant dans l'offre ? Monsieur le secrétaire d'État, comment prétendre vouloir réussir la transition écologique tout en permettant, sous couvert de décentralisation et par le jeu de la concurrence, la rétraction du réseau et la diminution de l'offre ? Comment le Gouvernement compte-t-il accompagner les régions pour garantir un haut niveau de service public, alors que la LOM n'a prévu aucune ressource nouvelle pour les autorités organisatrices ?

son système ferroviaire, ce qui n'est pas le cas chez nous, où le réseau reste bien un monopole national. La société SNCF demeure une société nationale à capitaux publics, qui, effectivement, est mise en concurrence sur le marché

en accordant des moyens considérables- 35 milliards d'euros de dettes repris, dont 25 milliards d'euros dès cette année -, ce qui permet à la fois de diminuer les frais financiers et de réinvestir massivement sur le réseau. J'ai donné les chiffres tout à l'heure. Vous parliez de moins-disant social. Je réponds que, avec l'ouverture à la concurrence, il est effectivement nécessaire de mettre en place des protections pour les salariés du rail à l'échelle de la branche. Tel est l'objet des discussions en cours pour la conclusion d'une convention collective de haut niveau. Ces travaux avancent bien et, autour de la mi-janvier, les principaux syndicats

ce cadre a permis, dans un certain nombre de pays- la Suède, l'Allemagne ... -d'offrir une offre de transport ferroviaire, notamment sur le TER, de meilleur niveau et à un coût plus acceptable pour l'usager et pour les collectivités publiques.

La grève entamée en décembre dernier est toujours d'actualité, et la prochaine ouverture à la concurrence inquiète. La question se pose d'autant plus que, en octobre dernier, la Cour des comptes s'interrogeait sur l'efficacité du modèle, notamment économique, des TER. Dans ma région, les Hauts-de-France, la nouvelle grille TER est entrée en fonction le 15 décembre dernier, mais l'évaluation des résultats est nécessairement retardée à cause des blocages que nous connaissons. J'ai cependant eu l'occasion, dès le 18 octobre, de saluer le cadencement renforcé entre la métropole lilloise et le Dunkerquois. Ce nouveau cadre est le fruit de négociations ardues entre la SNCF et le conseil régional ; il inclut une clause de rendez-vous essentielle. L'ambition politique collective est claire : la réussite des territoires et de la région. Le réseau TER constitue un pilier essentiel du dynamisme de nos régions et une source d'opportunités pour nos concitoyens. Une offre adaptée correspondant aux spécificités de chaque territoire est primordiale afin de répondre au mieux aux besoins des Français. La mise en concurrence apparaît, selon certains, comme une solution pour améliorer la qualité de l'offre TER dans nos régions, et garantir un service public ferroviaire efficient. À l'heure où les premiers appels d'offres de mise en concurrence voient le jour, notamment en région PACA, pensez-vous, monsieur le secrétaire d'État, que la SNCF, nos régions et, surtout, nos infrastructures soient prêtes à faire face à l'arrivée de la concurrence ? La parole

au gré des rencontres que j'ai pu avoir avec les syndicats du ferroviaire, en tout cas avec les syndicats progressistes, qui sont venus échanger avec nous, nous avons posé un certain nombre de garanties pour les cheminots, de même que pour les agents de la RATP. Ces éléments, qualifiés d'ailleurs par certains de bon compromis, permettent à la fois

Nous disposons en revanche, depuis octobre dernier, du rapport de la Cour des comptes sur « les transports express régionaux à l'heure de l'ouverture à la concurrence », dans lequel cette instance émet neuf recommandations. L'une d'entre elles a retenu mon attention, car elle formalise une vision que je défends depuis de nombreuses années, à savoir la nécessité de réaliser une analyse sociale, économique et environnementale de chaque ligne peu fréquentée, permettre à chaque région de choisir entre les options suivantes : développer la ligne ; la maintenir en la gérant de façon plus économique ; l'organiser avec un autre mode de transport, ce qui peut d'ailleurs induire un changement d'autorité organisatrice ; enfin, la supprimer. Sont concernées les régions, bien sûr, mais aussi SNCF Mobilités et SNCF Réseau. Je me permettrai de compléter cette recommandation en intégrant une option complémentaire, qui consiste à confier la ligne à un autre opérateur dans le cadre de l'ouverture à la concurrence, en associant dans le tour de table les collectivités locales et territoriales, ainsi que les intercommunalités, qui ont une place importante dans la LOM récemment promulguée, sans oublier la métropole de Lyon, collectivité locale de plein droit à statut particulier. Dès lors, ma question est simple

utilisés les articles de la LOM prévoyant notamment l'implantation ou l'expérimentation de solutions innovantes, comme le train léger ou le train hydrogène. Je le redis, c'est bien ce cadre complet qui est mis en place aujourd'hui. Le temps n'est plus aux rapports ; le temps est à l'action. Ces accords bilatéraux seront signés,

Monsieur le secrétaire d'État, depuis le 3 décembre dernier, en application du nouveau pacte ferroviaire, les régions ont la possibilité de signer des contrats de service public de transport ferroviaire de voyageurs avec des opérateurs autres que SNCF Mobilités. Il s'agit d'une réelle avancée pour ces collectivités, qui espèrent améliorer leur service régional de transport ferré et profiter d'une baisse des coûts de fonctionnement, aujourd'hui à leur charge. Un rapport récent de la Cour des comptes fait d'ailleurs état d'un fort investissement des régions dans ce domaine entre 2012 et 2017, avec 2,1 milliards d'euros investis sur le réseau et les gares. ce rapport rappellent aussi que la propriété du réseau et des gares relève non pas des régions, mais bien de SNCF Réseau et de SNCF Mobilités. Cela dit, j'aimerais m'attarder sur la situation particulière des petites lignes ferroviaires, qui d'un rapport du préfet Philizot, commandé par le Gouvernement, mais toujours pas rendu public. Ces petites lignes sont presque toutes menacées par défaut d'entretien. C'est notamment le cas dans ma région des Pays de la Loire. Or, nous sommes tous d'accord pour le dire ici, les plus petites lignes sont essentielles au développement équilibré de l'ensemble du territoire. Cela fait explicitement partie des objectifs de la LOM. Pour répondre en partie LOM. Pour répondre en partie à cette problématique, la Cour des comptes préconise de clarifier les rôles respectifs des régions, du groupe public ferroviaire et de l'État dans le financement des infrastructures. Elle va même plus loin en suggérant de transférer aux régions qui le souhaitent la propriété des infrastructures régionales et de leur laisser le choix des modalités de gestion et d'entretien. J'y vois, à titre personnel, une possibilité intéressante, notamment en ce qui concerne les petites gares locales, qui pourraient jouer le rôle de lieux multimodaux accueillant d'autres services publics ou privés. Monsieur le secrétaire d'État, une clarification du rôle de chacun dans l'entretien du réseau et des gares fera-t-elle partie de votre plan d'action pour les petites lignes ? Donneriez-vous des moyens financiers suffisants aux régions, qui en récupéreraient la responsabilité, dans le cadre des solutions innovantes que vous avez évoquées tout à l'heure ?

ou régionales à faible trafic peut être réalisé vers des autorités organisatrices du transport ferroviaire qui en feraient la demande, sous réserve de l'accord du ministre des transports. Ensuite, il permet à SNCF Réseau de mettre en place des partenariats publics-privés pour la régénération, puis l'entretien

c'est bien de voir l'État, SNCF Réseau, les régions se mettre d'accord sur une clé de financement, en fonction de la typologie des lignes concernées. J'ai parlé des lignes les plus structurantes, c'est-à-dire de celles qui sont très fréquentées, des lignes qui font déjà l'objet de CPER et des lignes qui, demain, feront l'objet, notamment au travers des dispositions de ces articles, de solutions innovantes.

Monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, dans un rapport publié le 23 octobre dernier, la Cour des comptes pointait la dégradation continue de la qualité de service des transports express régionaux. Les magistrats y dénonçaient, notamment, un sous-investissement récurrent dans les infrastructures. En France, l'âge moyen des voies est d'environ 30 ans, contre 17 ans chez nos voisins allemands. Le propriétaire chargé de leur entretien, SNCF Réseau, reconnaît que moins d'un tiers de ces lignes régionales sont en bon état. Cet état dégradé du réseau conduit à des retards, voire à des suppressions de train pour des raisons de sécurité. Par exemple, la région Pays de la Loire a choisi de privilégier le ferroviaire. L'offre s'est accrue de 23 % sur la période 2012-2017, mais la fréquentation a stagné, car la concurrence est vive entre les TGV et les TER pour circuler sur des infrastructures ferroviaires saturées. C'est d'ailleurs pour cette raison que trois liaisons quotidiennes viennent d'être supprimées entre Angers et Le Mans. Il existe une grande hétérogénéité dans la fréquentation des lignes. Certaines, autour des métropoles, sont surchargées et peuvent être inconfortables pour les voyageurs. D'autres concourent à l'aménagement du territoire et au désenclavement de zones rurales, avec des gares parfois peu fréquentées. Ces dernières, déjà fragilisées par leur vétusté, doivent subir, comme l'ensemble du réseau, une réduction du nombre de contrôleurs dans les trains et de nombreuses fermetures de guichets. Dans ces conditions, comment pouvoir offrir au public un égal accès à l'offre de mobilités ? L'ouverture à la concurrence, obligatoire dans toutes les régions en décembre 2023, pourrait constituer une menace fatale pour ces lignes, qui jouent un rôle considérable contre les fractures territoriales. Le Premier ministre a annoncé sa volonté d'investir 200 millions d'euros supplémentaires dans les infrastructures ferroviaires à partir de 2022, alors que, selon le préfet Philizot, lors de son audition par le Sénat, le besoin a été évalué à 7,4 milliards d'euros pour la seule remise en état du réseau des lignes de desserte fine du territoire.

secrétaire d'État. Monsieur le sénateur, vous avez parlé de sous-investissements chroniques sur le réseau, et vous avez parfaitement raison. Vous avez souligné que notre réseau a, en moyenne, 30 ans d'âge, mais parfois, sur certaines petites lignes, c'est plus de 80 ans qu'ont les plateformes et les voies.

éclairé par des plans d'action régionaux et supporté de façon partenariale par l'État, SNCF Réseau et les régions. C'est l'objet des discussions que j'ai pu avoir, fin décembre, avec

tout d'abord à remercier le groupe Les Républicains d'avoir programmé ce débat, tant il est vrai que la situation des transports express régionaux est pour le moins floue. La SNCF avait pourtant lancé en 2016 un plan stratégique, Cap TER 2020, orienté vers la réduction des coûts et l'amélioration de la qualité des TER,

Enfin, en octobre dernier, la Cour des comptes déplorait un état dégradé du réseau et un service insuffisant pour un transport coûteux. Où en est-on des efforts de transformation du TER en ce début d'année 2020, qui marque l'ouverture à la concurrence ? On le sait, deux chantiers sont prioritaires. Le premier est celui de la réorganisation des rôles respectifs des régions, du groupe public ferroviaire et de l'État dans le financement des infrastructures. Le second chantier de modernisation du TER est celui de son attractivité. Il doit être valorisé, car il constitue un mode de transport s'ancrant dans les territoires de nature à accompagner la transition énergétique.

Ainsi, la régularité du TER s'est améliorée, passant de 91 % sur les cinq premiers mois de 2017 à 93 % sur les mêmes mois en 2019, ce qui est tout à fait encourageant. Le trafic TER a augmenté de près de 4 % sur la même période. Les charges d'exploitation, en hausse continue depuis 2012, ont diminué entre 2017 et 2018.

Ligne à voie unique, sa rénovation, réclamée depuis plus de trente ans par la société civile et les élus locaux, a débuté en 2013 par la réfection complète de la section entre Dinan Cette même société civile, au travers d'une association et des élus locaux, a obtenu de haute lutte la poursuite de la rénovation entre Pleudihen-sur-Rance et Dol-de-Bretagne. Celle-ci a commencé en décembre 2019 et devrait durer une année. Elle permettra d'améliorer l'offre de transport entre Dinan et Rennes et entre Dinan et Saint-Malo. Ces travaux sont estimés à 62 millions d'euros et prévoient la rénovation de la section Dinan-Lamballe vers Saint-Brieuc. Inscrits au CPER 2015-2020, quelque 26 millions d'euros sur 62 millions concernent la première partie. Les 36 millions d'euros restants sont affectés à la rénovation de la section Dinan-Lamballe. Le calendrier n'étant pas encore bien établi, la société civile et les élus locaux craignent une rupture entre les travaux qui sont en cours et ceux de la partie occidentale de la ligne. pour la pérennité des financements qui ont été actés en 2015 et qui se terminent à la fin de cette année avec le contrat de plan. La continuité des travaux entre les deux parties de la ligne est indispensable. Les retards et tergiversations ont assez duré SNCF Réseau, seul maître d'oeuvre de ces rénovations, demande aux collectivités et à l'État de provisionner des montants considérables, aussi bien pour les études que pour les travaux, avec, monsieur le secrétaire d'État, un manque total de transparence sur les fonds publics versés par les collectivités à SNCF Réseau. Monsieur le secrétaire d'État, pouvez-vous m'assurer de la continuité des travaux et du maintien du fléchage des 62 millions d'euros, pour, enfin, finir la rénovation du barreau nord Côtes-d'Armor-Ille-et-Vilaine, tant attendu par les élus et nos concitoyens ?

le pacte d'accessibilité et de mobilité pour la Bretagne, le 8 février 2019, l'engagement de l'État sur les 5,6 millions d'euros qui ont été contractualisés pour garantir la convention de financement des travaux sur la section Dol-de-Bretagne-Pleudihen, que vous avez citée, et, au même titre que les partenaires du CPER, pour apporter les crédits nécessaires à la réalisation des travaux de la section Dinan-Lamballe, que vous avez également citée et dont les études se poursuivent jusqu'à la fin de 2020. Dans l'attente de ces prochains travaux, SNCF Réseau consacre depuis 2018 une somme de 350 000 euros par an à la maintenance renforcée pour garantir la circulation des trains et le déplacement des voyageurs. Je vous confirme que l'objectif est bien d'assurer la continuité de ces opérations entre les CPER, qui courent jusqu'en 2022, éventuellement à l'aide d'avenants, et la nouvelle génération des contrats, l'idée étant évidemment d'assurer la continuité du service public ferroviaire.

je me réjouis de ce débat, que l'on doit au groupe Les Républicains et qui porte sur un sujet du quotidien pour nos concitoyens, en particulier ceux qui vivent en périphérie des grandes métropoles ou des grandes agglomérations. Je regrette toutefois que ce débat soit limité à la seule question des TER. Il me semble en effet que, pour améliorer la mobilité de nos concitoyens, il faut penser intermodalité et non pas mode par mode. J'en viens à ma question. En octobre 2018, le P-DG de SNCF Réseau souhaitait sous-traiter certaines petites lignes au privé. Laisser le privé gérer la maintenance ou l'exploitation de certaines lignes était vu comme une solution pour augmenter leur rentabilité ; dans le cas contraire, la dette de SNCF Réseau allait se creuser. Des critiques avaient été émises sur les risques pour la sécurité du réseau

sur la sous-traitance privée de la maintenance ou de l'exploitation de certaines lignes de TER

Vous avez rappelé ce qui pourra être mis en oeuvre au travers des travaux de la mission Philizot. La région est tout à fait allante sur la ligne Nancy-Vittel pour mettre en oeuvre l'article 172 de la loi et ainsi trouver les voies de la pérennisation de cette ligne. C'est par ces efforts concertés, par l'activation de l'ensemble de ces dispositifs au bénéfice des petites lignes que nous arriverons

Le 10 mai dernier, la région a publié un avis de pré-information sur les services qu'elle entend réattribuer à compter du mois de mai 2020. Elle ne dispose plus que de six mois pour préparer les appels d'offres, et SNCF Voyageurs profite de sa situation de monopole en ne transmettant pas les informations nécessaires. Pourtant, la région a veillé à signaler son besoin avec un maximum d'anticipation. En effet, le 12 mars 2018, une première demande a été formulée par courrier. Au lendemain de la promulgation de la loi pour un nouveau pacte ferroviaire, la demande a été réitérée. Il convient de préciser que les dispositions concernant les informations dues aux autorités organisatrices par les opérateurs ferroviaires étaient pleinement applicables. Le 13 novembre 2018, la région Hauts-de-France a renouvelé et complété sa demande, après avoir rempli l'obligation préalable d'adopter un plan de gestion des informations couvertes par le secret des affaires, tel qu'en dispose la réglementation idoine, que l'État a mis plus d'un an à préciser dans un décret du 20 août 2019. Enfin, le 15 octobre dernier, dans un contexte d'information asymétrique dénoncé par la Cour des comptes et par la chambre régionale des comptes, la région a adopté un nouveau contrat de service public, sans pour autant avoir pu obtenir contractuellement les informations recherchées. Face à l'absence de transmission des informations de la part de l'opérateur historique, la région, dans l'incapacité d'exercer pleinement ses prérogatives, a saisi l'Autorité de régulation des transports (ART) dès le 19 avril 2019. À cette occasion, elle a pu préciser ses demandes d'information dans de nombreux courriers et au cours de cette procédure contentieuse. À ce jour, le règlement de différend n'a pas encore abouti, et l'acte de régulation sur lequel le collège de l'Autorité aura à se prononcer est, quel qu'en soit son contenu, susceptible d'un recours de SNCF Voyageurs, ce qui retarderait davantage la mise en oeuvre effective de la réforme voulue par le législateur. Il apparaît donc urgent

Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, le 4 décembre dernier, l'État et les collectivités locales ont annoncé, lors d'un comité interrégional, le financement de la rénovation de la ligne ferroviaire Grenoble-Veynes,

Lors de ce dernier comité de pilotage, SNCF Réseau a annoncé qu'une communication positive serait faite début 2020 pour valoriser l'engagement de l'ensemble des partenaires pour le maintien durable du service.

de rechange devenue de plus en plus fréquente hors période de travaux ; je ne dresserai pas ici la liste des exemples qui se multiplient, notamment dans mon département des Hautes-Alpes. Or le recours au transport par la route doit rester occasionnel, qui plus est sur les lignes régionales, où la tentation est grande de fermer les guichets, puis les gares et, demain, les lignes. raison pour laquelle, monsieur le secrétaire d'État, les élus, tant de l'Isère que des Hautes-Alpes, et les usagers ne peuvent se satisfaire des réponses techniques apportées aujourd'hui par SNCF Réseau et demandent à l'État de ne pas relâcher sa vigilance pour obtenir de l'exploitant le maintien des trajets intégralement en train, sauf en cas de force majeure.

En contrepartie de la prise en charge par l'État du renouvellement complet du matériel ferroviaire, la région s'est investie dans l'amélioration des transports du quotidien par sa gouvernante. Grâce à ses choix, les usagers des lignes Paris-Caen-Cherbourg et Paris-Rouen-Le Havre embarqueront bientôt dans des

de la régénération des voies. La région Normandie a évidemment fait valoir ses besoins. Elle participera de la même façon aux accords bilatéraux que nous envisageons de signer de façon tripartite avec SNCF Réseau, de manière à faire plein usage de l'article 172 de la loi d'orientation des mobilités et de permettre,

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, le Sénat ne perd jamais une occasion de parler de la ruralité. Tout d'abord, parce que le Sénat « assure la représentation des collectivités territoriales de la République » et que celles-ci sont rurales à 90 %. et surtout, parce que les élus locaux savent à quel point les maux dont souffre le monde rural sont profonds. Et ses habitants vivent avec le sentiment d'évoluer dans une société bloquée, qui entrave la promesse républicaine d'égalité.

Néanmoins, la réforme de 1963 n'a pas consisté en la création d'une nouvelle direction hyperspécialisée : elle a reposé sur un objectif simple, à savoir créer des pôles de croissance capables de réorienter les flux économiques avec un pilotage pragmatique et, surtout, des moyens financiers. Très exactement le contraire de la situation actuelle ! Cette politique a fonctionné aussi longtemps qu'elle a été maintenue. Hélas, les chocs pétroliers et leurs conséquences auront peu à peu conduit à considérer l'aménagement du territoire comme un luxe superflu. la ruralité n'a droit qu'à des soins palliatifs. Un bel exemple : on veut recréer des cafés, des stations-service, des petits commerces et redynamiser les bourgs-centres, après avoir tout fait pour les faire disparaître avec, entre autres, de gigantesques zones commerciales. C'est donner un cachet d'aspirine à quelqu'un sur qui on a tiré au bazooka ! Aujourd'hui, en 2020, le volume total des dispositifs d'aide est au plus bas. Je vous renvoie à la lecture du rapport de mon collègue Louis-Jean de Nicolaÿ sur le budget 2020, qui détaille les crédits consacrés à l'aménagement du territoire.

Certains pensent encore que l'économie numérique va créer un mouvement massif et spontané vers le monde rural, qu'une start-up corrézienne ou, mieux, ardéchoise pourra travailler sans difficulté avec des clients brésiliens et des fournisseurs coréens. jusqu'à présent, le développement du numérique a encore accentué la concentration géographique de la création de richesses. Je pense, par exemple, à l'installation de la fibre optique, gratuite pour les grandes agglomérations et payante pour les autres territoires. Ainsi, la communauté de communes de la Montagne d'Ardèche, avec ses 5 000 habitants, devra payer 2 millions d'euros. Quel bel exemple de solidarité territoriale Avant d'espérer, il faut déjà s'accorder sur certains postulats et tailler en pièces les idées reçues : oui, le monde rural peut s'insérer dans la mondialisation ; oui, le monde rural peut accueillir des activités économiques à forte valeur ajoutée ; enfin, non, le monde rural ne peut être cantonné au rôle de réserve naturelle destinée à combler la soif d'authenticité de nos amis citadins. Concrètement, nous connaissons les deux défis à relever l'un est économique, l'autre démographique. Aujourd'hui encore, les jeunes quittent le monde rural par manque de débouchés, et les entreprises ne s'y installent pas, faute de main-d'oeuvre. Il existe, madame la ministre, beaucoup de propositions intéressantes dans le plan du Gouvernement, et parfois des propositions de bon sens, qui ne sont ni coûteuses ni complexes à mettre en oeuvre. Vous savez pourtant, madame la ministre, que deux difficultés majeures préoccupent les élus que nous sommes : la fracture numérique et les déserts médicaux.

Pis encore, comment voulez-vous y retenir des habitants qui perdent patience ? Cela n'a rien d'étonnant : quand on prend conscience que l'on n'a accès ni aux mêmes droits ni aux mêmes chances que ses compatriotes, l'impatience se transforme en colère. La révolte des « gilets jaunes » s'illustre ainsi par quatre revendications essentielles : ils veulent pouvoir nourrir leur famille, se loger décemment, se déplacer et, surtout, se faire soigner. Le reste n'est que littérature

renforcer le champ d'intervention des professionnels de santé non-médecins et d'assurer le déploiement de 400 postes de médecins salariés. Si l'on ne peut que soutenir ces mesures, je rappelle qu'elles sont de court terme, et que leur dose n'est qu'homéopathique. S'agissant des réponses à plus long terme, vous proposez de déployer les stages d'internes en médecine dans les zones sous-denses, en priorité dans les territoires ruraux. Nous souscrivons évidemment à cette proposition

J'irai jusqu'à dire qu'il y a une certaine indécence à produire un plan d'action aussi ambitieux pour, à peine trois mois plus tard, soumettre à consultation un nouveau cahier des charges pour le financement des réseaux d'initiative publique qui conduira, tout simplement, à la disparition du plan France très haut débit. Les habitants du monde rural- vous le savez, madame la ministre -n'attendent pas de miracles. À force de promesses non tenues, ils sont devenus indifférents aux grandes opérations de communication dont ils sont les

qui peut nous laisser penser que cette initiative aura un sort différent de celui des comités interministériels aux ruralités, lancés par la précédente majorité, où de vos conférences territoriales, déjà oubliées ? Mobilité, santé, emploi, accès aux nouvelles technologies : souvenons-nous que le monde rural et les ruralités sont au carrefour de toutes les grandes problématiques du XXI siècle. Y répondre, c'est déjà préparer, pour tous les Français, l'émergence d'une nouvelle société au sein de laquelle le monde rural aura davantage qu'une place : un avenir ! La parole

visait à dresser le bilan des dispositifs de soutien aux territoires ruraux les plus fragiles. Plus récemment encore, la délégation aux collectivités territoriales de la Haute Assemblée a organisé un colloque sur le rôle des collectivités territoriales comme levier de développement pour la ruralité.

que j'ai mis en place une mission composée d'élus ruraux. J'ai souhaité m'appuyer sur leur expérience et sur leurs propositions, avec l'objectif, à la fois simple et complexe, d'améliorer la vie quotidienne des habitants des territoires ruraux. Après plusieurs mois de travaux, ces élus m'ont remis un rapport où figuraient 200 propositions. Le Gouvernement s'est appuyé sur ces recommandations pour élaborer l'agenda rural annoncé par le Premier ministre le 20 septembre dernier à l'occasion du congrès de l'AMRF à Eppe-Sauvage, dans le Nord. Mesdames, messieurs les sénateurs, cet agenda rural est le premier plan d'action mené par un gouvernement en faveur des ruralités à regrouper des enjeux aussi larges que la transition écologique, l'agriculture, l'éducation, la santé, la formation, l'emploi, le développement économique et la culture. Plus encore,

Cet agenda constitue désormais le cadre gouvernemental de mise en oeuvre des politiques publiques d'aujourd'hui et de demain en faveur des territoires ruraux. S'il comporte à ce jour 181 mesures,

De manière inédite, j'ai souhaité y associer les auteurs du rapport de la mission « Agenda rural », tant parlementaires que représentants des associations d'élus, qui pourront ainsi suivre la mise en oeuvre complète de ce plan d'action. Depuis le 1 janvier, plusieurs dispositifs de l'agenda rural sont d'ores et déjà effectifs. Il s'agit, notamment,

Nous avons souhaité déployer ce nouveau réseau pour offrir aux habitants de ces territoires un service public de proximité et de qualité. Nous avions tous fait le constat que les services publics avaient beaucoup reculé sur nos territoires.

Requier. Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, je tiens à saluer, en préambule, la création au 1 janvier 2020 de l'Agence nationale de la cohésion des territoires, portée par notre groupe, qui devrait être fortement mobilisée dans le cadre de l'agenda rural pour accompagner les projets portés par les élus locaux, au travers d'un soutien en ingénierie et de la prise en compte de leurs spécificités. Nos territoires ont un potentiel d'attractivité inexploité. Tel est le cas des petites villes, dont un regain d'activité peut avoir un effet particulièrement bénéfique pour les territoires ruraux environnants. Au-delà de l'amélioration de l'habitat et du cadre de vie, il est impératif de favoriser le retour de la vie économique et de l'emploi dans ces petites villes. N'oublions pas d'encourager la renaissance des petits commerces, des cafés et des bistrots, des bistrots, lieux de vie et de convivialité qui disparaissent ! Sans de tels efforts, le bâti sera certes agréable, mais il restera vide ! L'ANCT pilotera cette année son premier programme territorialisé : le plan Petites villes de demain, annoncé en septembre dernier. Il s'agira, je l'espère, d'une concrétisation de l'utilité de cette agence, mais aussi d'un changement de logique et de culture administrative. Les élus doivent être associés à l'élaboration de cette politique publique. Entre 800 et 1 000 villes de moins de 20 000 habitants exerçant une fonction de centralité devraient être sélectionnées en fonction du nombre et de la nature des équipements dont elles disposent, ainsi que sur des critères de fragilité. Un indice lié à l'éloignement, qui permet de mesurer le temps d'accès au prochain pôle de centralité, mesure pourtant essentielle, ne serait utilisé qu'en dernier recours, à la lecture de l'instruction adressée aux préfets. Madame la ministre, pourriez-vous nous préciser la pondération des critères retenus pour la sélection des villes concernées, afin de garantir un ciblage des territoires les les plus fragiles, ainsi que les moyens financiers consacrés à cette initiative

à hauteur de 25 % et prendra en charge à 100 % les missions d'assistance au management de projet pour les territoires en difficulté. Par ailleurs, elle interviendra au travers de l'octroi de prêts et investira dans certains projets.

le plan d'action en faveur des territoires ruraux présenté en septembre dernier traduit l'ambition forte du Gouvernement en faveur de la cohésion territoriale et de la lutte contre les inégalités et les disparités entre zones rurales. Par cet agenda rural,

dans le rapport sénatorial sur la revitalisation des centres-villes et centres-bourgs. L'un des axes principaux du plan d'action en faveur des territoires ruraux est le soutien aux petits commerces et aux lieux de convivialité. Est notamment prévu un appui de votre ministère à l'initiative « 1 000 cafés », qui est portée par le groupe SOS, acteur essentiel de l'économie sociale et solidaire. Il s'agit de revitaliser les communes rurales, en ouvrant ou en reprenant 1 000 cafés dans 1 000 communes de moins de 3 500 habitants n'ayant plus de café ou risquant de les perdre. Les appels à candidatures à destination des maires ont été lancés le 12 septembre 2019.

élus ? Comment vos services travaillent-ils concrètement avec le groupe SOS pour superviser cette action essentielle au renforcement sinon au maintien du lien social en milieu rural ? La parole

ne disposent plus de cafés ou dont le café subsistant voit sa survie menacée. Depuis le lancement de cet appel à candidatures, le groupe SOS a reçu 500 candidatures de communes souhaitant accueillir un café sur leur territoire et 1 200 candidatures spontanées de personnes souhaitant

et démocratique qui est au coeur de mon engagement politique. Lutter contre l'artificialisation des sols, promouvoir l'agroécologie, faire des forêts le poumon de notre pays, revitaliser les petites villes, soutenir le commerce de proximité, lutter contre les déserts médicaux, faciliter l'accès aux services publics, développer l'ingénierie publique : à part le développement à l'aveuglette de la 5G, vous feriez presque carton plein ! Je parle au conditionnel, parce que, malheureusement, comme d'habitude, ce travail relève de l'opération de communication. Concrètement, vous ne mettez pas un euro sur la table. En outre, vos propositions vont souvent à l'encontre de la politique de votre gouvernement. Ainsi, vous voulez développer l'agroécologie tout en supprimant les aides au bio, préserver nos forêts tout en démantelant l'ONF, l'Office national des forêts, soutenir le commerce de proximité tout en permettant aux grandes surfaces de consigner le plastique, lutter contre les déserts médicaux sans contraindre, même, les médecins,

notamment dans le domaine de la mobilité, enjeu prioritaire pour nos concitoyens. Les territoires ruraux n'ont pas besoin de lignes aériennes subventionnées qui les mettraient à une heure de Paris ; ils ont besoin de dessertes ferroviaires fines, dont le sort est à nouveau renvoyé au rapport Philizot, l'on attend comme on attend Godot ; ils ont besoin de transports publics structurants qui permettent la mise en place de solutions adaptées à chaque contexte- covoiturage, vélo électrique, autopartage -, de manière à limiter l'usage de la voiture individuelle ; ils ont besoin que l'on parle, enfin, de « démobilité » et d'un aménagement du territoire équilibré, qui reviendrait sur l'hypermétropolisation,

l'artisanat et le commerce (Fisac) a su s'imposer comme un formidable levier de développement de l'attractivité et du dynamisme économique des territoires, en contribuant au maintien du tissu économique local. Ce fonds joue un rôle essentiel pour la revitalisation du commerce et de l'artisanat sur l'ensemble du territoire. Il constitue donc un instrument de développement local très important, puisqu'il a financé jusqu'à 1 000 projets annuels de soutien, de revitalisation, ou de reprise d'entreprises commerciales et artisanales de proximité. Malgré son efficacité, le Fisac a vu sa dotation passer de 78 millions d'euros en 2010 à seulement 16 millions en 2018. Depuis 2019, ce fonds est placé en gestion extinctive,

et non des bourgs en zones rurales, et, d'autre part, il ne cible pas tout à fait les mêmes actions. Force est de constater que ce dispositif est moins souple et moins adaptable aux spécificités locales.

Madame la ministre, pouvez-vous nous préciser quelle solution vous comptez promouvoir dans votre plan d'action, afin de poursuivre l'accompagnement et le maintien de nos entreprises de proximité, notamment en milieu rural ?

adoptée dans le cadre de la loi de finances pour 2020 et elle est effective depuis le 1 janvier. Elle consiste en la possibilité d'ouvrir, pour les collectivités qui le souhaitent, des zones de revitalisation commerciale qui permettent de bénéficier d'exonérations fiscales sur la cotisation foncière

que les territoires puissent se saisir de cette nouvelle opportunité en faveur du soutien aux petits commerces dans nos campagnes.

À mon sens, le point premier de toute politique à destination des territoires ruraux doit traiter du sujet vital, essentiel et primordial qu'est la santé. En effet, qui viendrait vivre dans une région, fût-elle la plus belle, la plus attractive, la plus charmante, offrant des possibilités d'accès à l'enseignement supérieur, au sport ou à la culture, s'il ne peut accéder aux soins ? Dans le chapitre du plan relatif à la santé, je lis en particulier qu'est prévue l'obligation pour les internes en médecine de réaliser un stage en zone sous-dense. Je me souviens même avoir voté au printemps dernier l'obligation pour les étudiants en fin de cycle de formation d'effectuer quelques mois d'exercice en zone déficitaire. À ce jour, cette mesure, qui serait pourtant une réelle avancée, attend son décret d'application. pour les mesures de délégation d'actes et de pratique avancée qui figurent dans le plan. De nombreux décrets d'application restent en attente : la liste des pathologies pour lesquelles les infirmiers pourront adapter la posologie de certains traitements, les modalités selon lesquelles les pharmaciens seront habilités à délivrer des médicaments pour certaines pathologies, les autorisations de vaccination des femmes et des enfants par les sages-femmes, la prescription par les pharmaciens de certains vaccins, la mise en oeuvre et les conditions de prise en charge des activités de télésoins, etc. etc. Madame la ministre, face à des enjeux cruciaux d'accès aux soins en milieu rural, sera-t-il possible de passer outre les pressions des différents professionnels et de mettre en application dans les meilleurs délais les mesures votées par le Parlement au mois de juillet dernier

Toutefois, le Gouvernement a souhaité anticiper ces échéances. L'un des facteurs limitants est le nombre de maîtres de stage accueillant des internes, malgré une hausse de 15 % en un an. Il faut donc aussi travailler sur ce sujet. viens aux nouvelles compétences des professionnels de santé. Dans le cadre des campagnes de vaccination hivernale, les pharmaciens peuvent désormais vacciner

effet, dans ce plan, on parle beaucoup de la médecine dite « de ville », mais pas de l'organisation des plateaux techniques chirurgicaux, publics ou privés. Dans le département de la Nièvre, dont je suis élue, il serait question d'un maillage terriblement large : rien entre Nevers et Montargis ou entre Bourges et Auxerre pour les urgences chirurgicales de nuit en faveur des territoires ruraux, vous comprendrez que cette situation n'est pas acceptable. Les déclarations et les actes sont par trop discordants. C'est pourquoi, madame la ministre, il faudrait traiter ces sujets, essentiels pour nous,

La voiture est aujourd'hui le moyen indispensable pour se déplacer dans les territoires ruraux ; je ne puis donc que saluer les mesures visant à permettre un accès plus rapide au permis de conduire, notamment grâce au développement des simulateurs de conduite et au permis à un euro par jour. qui contenait également des dispositions permettant, entre autres, à La Poste d'accueillir des élèves. Toutefois, il est important que nos concitoyens qui ont choisi de vivre ou de s'installer dans les territoires ruraux puissent eux aussi avoir accès à une offre de mobilité pertinente et adaptée à la situation locale. Le Sénat a oeuvré pour faire de la loi d'orientation des mobilités un véritable texte de lutte contre les zones blanches de mobilité. Ainsi, les intercommunalités pourront, si elles le souhaitent, organiser leurs propres solutions de mobilité dans leur territoire, afin de permettre à nos concitoyens d'avoir accès à cette intermodalité.

Sans ces moyens financiers, ces évolutions législatives n'auront pas de portée suffisante. Madame la ministre, que comptez-vous proposer pour répondre aux attentes légitimes sur ce sujet, dans l'intérêt de nos concitoyens

de la compétence mobilité dans la ruralité. Plusieurs solutions sont envisageables. Évidemment, il a été discuté- je mets à ce terme tous les guillemets qui s'imposent -de créer le versement transport

On peut néanmoins déplorer un grand manque de précisions, tant sur la question du financement que sur celle du calendrier des actions proposées. De nombreux sujets sont évoqués, et je pourrais m'attarder sur les propositions concernant la revitalisation des petites villes, qui pèchent par leur imprécision et leur incohérence. S'il est louable de souhaiter revitaliser les centres-bourgs, pourquoi alors avoir supprimé le Fisac il y a un an ? Je m'attacherai à évoquer seulement deux points, qui préoccupent particulièrement nos territoires. Sur le déploiement de la 5G, votre plan d'action s'occupe des détails avant de se concentrer sur l'essentiel. « Résorber les zones blanches pour renforcer l'attractivité des territoires » et équiper tous les pylônes existants en 4G d'ici à la fin 2020 ne répond absolument pas à la problématique des zones dites « grises ces zones couvertes par un seul opérateur, ni à celle des zones où les réseaux sont défaillants et où les pannes d'internet et la baisse des débits sont fréquentes. Cela concerne de nombreux territoires ruraux et montagnards, où les habitants ressentent une forme d'insécurité, mais avant tout un sentiment d'abandon et de fracture numérique. De même, sur le maillage territorial des services publics, vous promettez une maison France services par canton d'ici à deux ans, mais les agents d'accueil seront rémunérés par les collectivités et le fonctionnement sera compensé par une dotation de l'État jusqu'à une date indéterminée. C'est particulièrement flou et inquiétant pour les collectivités, qui voient leurs charges et leurs missions s'alourdir. Cette proposition suit exactement la même problématique que celle de la modernisation des services des trésoreries, où l'État prévoit d'augmenter les accueils de proximité, qui seront en réalité de simples permanences de conseil, sans possibilité de transactions, et où très peu de services seront proposés. Le tout-numérique ne peut pas être la seule solution aux besoins de proximité de nos territoires ruraux. Votre plan, qui se veut une réponse aux légitimes inquiétudes des élus locaux et des habitants, est flou, ce qui ne tend pas à les rassurer.

souvent, les collectivités territoriales, les régions, les départements, les intercommunalités, les communes participent à un certain nombre de financements. La réponse aux

qui sont à l'initiative de cette politique ; dans d'autres, ce sont des syndicats, qui existent dans les départements ou sur deux départements. Ce sont des politiques que nous contractualisons

la question de la santé et de l'accès aux soins médicaux est arrivée en tête des préoccupations. En effet, 4 millions de Français vivent dans des territoires en situation alarmante en matière d'accès à des professionnels de santé. Cette situation très grave est particulièrement difficile à vivre pour nos concitoyens habitant dans des territoires ruraux, déjà fortement touchés par la fracture territoriale. Le plan d'action en faveur des territoires ruraux comprend un volet consacré à la question des déserts Face à cette urgence, le plan propose notamment le recrutement de 600 médecins salariés dans les zones à faible densité, le déploiement de médecins supplémentaires et d'internes dans ces zones. Ce sont des mesures nécessaires, mais largement insuffisantes. L'un des objectifs de votre plan d'action est de soutenir les initiatives locales dans les campagnes. Précisément, en matière de santé et d'accès aux soins, des initiatives locales efficaces existent et méritent d'être mieux mises en valeur. Je pense en particulier au dispositif PAIS, plateforme alternative d'innovation en santé, qui est et que vous connaissez bien, madame la ministre. Le dispositif PAIS revitalise l'offre de médecine de proximité en favorisant les synergies entre médecins, au sein d'un même bassin de vie. Cela passe, par exemple, par la mutualisation du secrétariat ou par l'organisation à tour de rôle de la prise en charge des soins sans rendez-vous. Depuis plusieurs années, PAIS fait ses preuves ! Cette forme d'organisation plus souple semble bien adaptée aux nouvelles pratiques des médecins généralistes de proximité. Le Gouvernement est-il disposé, avec l'appui des médecins qui le souhaitent, à faire entrer ce dispositif dans les mesures de soutien à la ruralité et, ainsi, à le généraliser à l'échelle nationale ? Et si oui, à quelle échéance ? La parole est à Mme la ministre.

dans son volet de stage à caractère éducatif, plus communément appelé « dispositif Argent de poche ». De nombreuses communes rurales ont mis en place ce dispositif permettant à des jeunes de travailler dans les collectivités territoriales ou dans des associations, jusqu'à ce que des préfets- comme cela a été le cas en Bretagne -, se réveillent et fassent valoir que ce dispositif n'était applicable que dans les quartiers dits « politique de la ville Je trouve cela fâcheux. Je sais que vous avez déjà été alertée sur ce sujet et que vous avez laissé espérer un réexamen de cette question, considérant qu'il n'y avait pas de raison que les jeunes ruraux ne puissent pas bénéficier de ce dispositif, d'autant qu'il semble

En 2015, les sommes versées aux jeunes âgés de 14 ans à moins de 26 ans, au titre de leur activité dans le cadre de ce programme, sont devenues assimilables à des gratifications versées aux stagiaires en entreprise. Elles sont par conséquent exclues de l'assiette des cotisations et contributions sociales dans les mêmes conditions. Si ce dispositif était initialement et est encore conçu seulement pour la politique de la ville, je sais que certains territoires, notamment en Bretagne, en particulier en Ille-et-Vilaine,

Cependant, si cela existe dans certains territoires, ce n'est pas le cas à l'échelon national et l'Association des maires ruraux de France (AMRF) a d'ailleurs récemment interpellé mes équipes à ce sujet. Dans ce cadre, j'ai souhaité solliciter ma collègue ministre de la santé, pour étudier les conditions d'une extension de ce dispositif aux territoires ruraux. Des échanges sont en cours. Je ne manquerai pas de vous tenir informé, tout comme l'AMRF d'ailleurs, de la suite que nous pourrons réserver à cette demande, qui me semble tout à fait légitime.

est à M. Hervé Gillé. Madame la ministre, un plan d'action et un agenda rural en faveur des territoires ruraux, oui, c'est incontournable : plus de 22 millions de Français vivent dans ces territoires, où s'additionnent les difficultés de mobilité et d'accès à l'emploi, aux services, à la santé. Dans le même temps, 22 métropoles capitalisent l'essentiel des richesses, des créations d'emploi, de l'accès aux mobilités, à la culture, à la santé ... Ces dynamiques métropolitaines s'accélèrent, et leur développement devrait bénéficier aussi aux villes moyennes, aux zones périurbaines et rurales. Ces métropoles fournissent des emplois, des services et des équipements qui profitent à la plupart, mais est-ce suffisant quand persistent autant d'inégalités territoriales ? L'opposition permanente entre métropoles et territoires ruraux ne peut être une fatalité ou une instrumentalisation politique. Nous voulons construire une alliance en complémentarité, mais il faut de nouvelles solidarités territoriales, des moyens concrets, un partage des richesses plus juste, un devoir vis-à-vis de territoires souvent déshérités, mais indispensables à nos équilibres. Ces territoires sont également des acteurs incontournables de la mise en oeuvre des politiques liées aux défis environnementaux ils constituent souvent les espaces de compensation nécessaires à l'activité urbaine, insuffisamment valorisés. Grâce à une forte concentration d'entreprises, les métropoles capitalisent des recettes fiscales, qui pourraient être des outils au service de contrats de coopération, dont la réciprocité financière n'est pas toujours assurée. Des propositions ont été formulées pour de nouvelles coopérations financières par des dispositifs de solidarité fiscale. Ainsi, le 1 % métropole, construit à partir des recettes de la contribution économique territoriale, n'aurait pas d'impact à l'échelle des métropoles, tout en offrant des perspectives.

La mesure de votre plan consistant à augmenter les ressources des autorités organisatrices des mobilités par une fraction de la TVA est insuffisante et, surtout, trop conjoncturelle.

entre les territoires. Nous ne pouvons qu'encourager ces dispositifs qui commencent à exister, mais qu'il faut améliorer, et que l'on appelle les contrats de réciprocité.

Louault, sénateur d'Indre-et-Loire. Lui aussi a mis en place des contrats de réciprocité. Aujourd'hui, ces contrats de réciprocité sont à la main entière des collectivités territoriales, sans cadre et sans incitation au partage de la ressource. Je le répète : il serait intéressant d'encourager ce dispositif de contrats de réciprocité et d'y réfléchir dans le cadre de la loi 3D.

je ne puis que souscrire à votre plan d'action en faveur des territoires ruraux. Les intentions sont belles et devront se traduire par des mesures concrètes. Rappelons nos atouts et les enjeux. Nos territoires constituent un véritable capital et représentent une formidable richesse. Nos campagnes doivent donc être un moteur du modèle écologique. La France, qui compte 30 000 millions d'hectares de surfaces agricoles, reste la première puissance agricole de l'Union européenne. L'agriculture est au coeur de la lutte contre le changement climatique. Elle en est l'une des principales causes, car le secteur agricole émet trop de gaz à effet de serre, mais elle en subit également les conséquences : sécheresses, inondations. À cela s'ajoutent les effets délétères du recours aux produits phytosanitaires sur les espèces et sur notre santé. L'agroécologie est la réponse

Il est donc urgent de soutenir nos agriculteurs et de leur apporter de véritables garanties financières, afin de leur permettre de modifier leurs pratiques. Nos systèmes de production doivent, plus que jamais, s'appuyer sur les potentialités offertes par les écosystèmes,

en développant, par exemple, les projets alimentaires territoriaux et les programmes agricoles expérimentaux. Ces projets fédèrent les acteurs d'un d'un territoire autour d'une ambition partagée pour développer l'agriculture durable et une alimentation de qualité. L'agenda rural prévoit également d'encourager l'approvisionnement en circuits courts des collectivités territoriales et des services déconcentrés de l'État ; c'est très important.

soutenir les nouvelles pratiques agricoles, notamment l'agriculture biologique et l'exercice collectif. Les initiatives vertueuses en matière d'écologie, les groupements d'intérêt économique et environnemental ou le volet agricole du grand plan d'investissement,

L'intensité des manifestations des « gilets jaunes », particulièrement fortes dans le Lot-et-Garonne, nous oblige à agir. Ayant été maire pendant vingt-cinq ans et infirmière libérale, je tenais à attirer votre attention sur les enjeux de démographie médicale et d'accès aux soins. Vous le savez, la situation s'est considérablement dégradée. Les collectivités locales ont pourtant pris leurs responsabilités en créant des maisons de santé ou en salariant des médecins, afin que ce service public vital ne disparaisse pas totalement de leurs territoires. du système de santé a permis de donner un souffle nouveau, en encourageant l'installation des médecins dans les zones sous-denses. Pour sa part, le Sénat a soutenu la pratique des délégations de tâches entre professionnels de santé, afin de faciliter l'accès aux soins.

Chaque année, 120 000 infirmiers libéraux interviennent auprès de 11 millions de patients, soit 18 % de la population, dans 90 % des cas à domicile. De même, 1,5 million d'aides à domicile interviennent auprès de plus de 3 millions de Français.

La multiplication des lotissements autour de nos beaux villages de Provence, ainsi que leur densification excessive, dénature leur authenticité et réduit leur attrait touristique. On ne peut plus tolérer aux abords des magnifiques villages du Lubéron ou du Ventoux la même densité de construction que dans les banlieues de nos villes, c'est une évidence.

Toutefois, le diable se cache souvent dans les détails. Vous proposez de permettre le recrutement mutualisé d'éducateurs sportifs polyvalents entre une commune ou une intercommunalité rurale et les acteurs de l'économie sociale et solidaire. Vous proposez également de renforcer le soutien aux clubs sportifs en milieu rural, notamment le soutien aux équipements sportifs et aux associations en milieu rural. vous souhaitez donc encourager les communes rurales à recruter du personnel qualifié. Malheureusement, nous savons tous que nombre d'entre elles connaissent de graves difficultés budgétaires, qui empêchent toute nouvelle dépense de fonctionnement. Quel soutien financier l'État compte-t-il apporter à

Madame la ministre, le développement de la pratique sportive dans nos territoires est une nécessité, alors que la sédentarité est une problématique très lourde pour les générations futures. D'autres propositions ont été formulées par les parlementaires, notamment ici au Sénat : soutien au mécénat, 1 % artistique et sportif, simplification des réglementations, développement de la pratique du sport à l'école. Quand le Gouvernement reprendra-t-il ces propositions ? Monsieur le sénateur, sachant que vous alliez m'interroger sur ce sujet, j'ai demandé à la ministre des sports de me donner quelques chiffres.

49 millions d'euros seront affectés au soutien de 4 151 emplois d'éducateurs sportifs au sein des clubs. Il a été demandé aux délégués territoriaux de l'Agence de veiller à accompagner le recrutement des emplois

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, nous achevons ce nouveau débat sur la ruralité. Assurément, ce ne sera pas le dernier,

c'est que nous sommes, aux termes de l'article 24 de la Constitution, les représentants des collectivités territoriales de la République et, de ce fait, les obligés, en quelque sorte, des élus locaux. La seconde, c'est que le Gouvernement n'a cessé, depuis sa formation, de renouveler les témoignages d'amour, de compassion et de considération à l'endroit des territoires ruraux, que je ne crois pas encore perdus. En politique, nous connaissions l'existence des « candidatures de témoignage ». Prenez garde de ne pas créer le concept de « politique publique de témoignage Les conférences des territoires ont laissé un goût amer à de nombreux élus, leur déception étant proportionnelle à l'enthousiasme que vous avez suscité chez eux.

qui est une émanation du rapport du 26 juillet 2019 de la mission « Agenda rural », dont l'AMRF était membre. Comme certains, je salue de bonnes idées et l'important Pourtant, je ne puis m'empêcher de relever une certaine dissonance entre ce plan, qui se veut la vitrine de votre politique publique en faveur de la ruralité, et vos actes quotidiens. J'aborderai en premier lieu les maisons France services. Évoquées par le Président de la République lors du grand débat national, ces structures doivent rapprocher les citoyens des services publics dont ils sont bénéficiaires. Comment s'opposer à une étant, plus le temps passe, plus je me demande si ces structures vont réellement apporter une valeur ajoutée par rapport aux actuelles maisons de services au public (MSAP). J'en viens même à me demander si elles ne constituent pas une régression déguisée. déguisée. Ces maisons vont-elles conserver une dimension véritablement rurale ? Surtout, pourquoi, comme nous le voyons aujourd'hui, adopter une approche technocratique de ces structures en les obligeant, par exemple, à disposer de deux équivalents temps plein ? Ceux qui se plaignaient du manque de souplesse des MSAP vont être servis avec les nouvelles maisons France services ! Je m'arrêterai en second lieu un instant sur le sort que vous réservez au plan France très haut débit.

C'est pour cette raison que le Sénat a souhaité, dans sa sagesse, amender la loi de finances, pour alimenter ce plan non pas en crédits de paiement, mais en autorisations d'engagement. Comme vous le savez, ce plan est le moteur de l'aménagement numérique de nos territoires. Avec cette décision, avec ce nouveau cahier des charges, vous actez la mort du plan France très haut débit. Dans un récent communiqué, vous avez d'ailleurs évoqué l'objectif de couvrir 92 % de la population, laissant 5,5 millions d'habitants sur le bord de la route.

L'ordre du jour appelle le débat sur la réforme des retraites,

dans quinze jours. Mais cela fait déjà plus d'un mois qu'a commencé un mouvement social d'ampleur, et cela fait plus longtemps encore que, bien au-delà des syndicats et des grévistes, les Français se posent des questions sur l'avenir de leurs retraites. C'est pourquoi, monsieur le secrétaire d'État, la commission des affaires sociales a souhaité l'organisation de ce débat au Sénat dès la rentrée, afin que le Parlement et, à travers lui, le plus grand nombre de nos compatriotes puissent dès à présent y voir clair sur l'essentiel. Qu'elle s'inscrive dans le présent, dans un proche avenir ou dans une perspective lointaine, chacun se sent concerné par la retraite. De ce fait, il s'agit d'un sujet politique hautement inflammable. Pour qu'une réforme, un changement complet des règles de calcul, soit acceptable, il faut que les Français aient confiance dans ce qui leur est proposé. Or on ne peut que constater qu'ils ne font guère confiance au Gouvernement. Pour partie, cette situation s'inscrit dans une évolution générale et préoccupante de défiance dans la parole publique. Mais, pour partie également, elle résulte directement des actions du Gouvernement, que le Sénat a régulièrement dénoncées.

le Gouvernement ne cesse de fouler aux pieds l'actuelle règle de revalorisation censée garantir que les pensions progressent au même rythme que l'inflation ? Gel des pensions en 2018,

000 euros : le Gouvernement a tout fait pour démonétiser sa propre parole et celle de ses successeurs. Par ailleurs, comment faire partager l'idée de travailler plus longtemps quand le Président de la République, durant sa campagne, n'a cessé de répéter qu'il ne toucherait pas à l'âge légal de départ à la retraite, sans jamais évoquer un quelconque âge pivot, quand ce même président clamait haut et fort son refus des réformes paramétriques et quand, depuis trois ans, vous n'avez cessé de vous opposer aux initiatives du Sénat visant à augmenter progressivement l'âge légal de départ à la retraite ? Comment les Français pourraient-ils s'y retrouver après de telles incohérences et un tel manque de pédagogie ? Enfin, comment nos concitoyens pourraient-ils croire à l'impérieuse nécessité de redresser les comptes de la branche vieillesse alors que, depuis deux ans, le Gouvernement a artificiellement réduit de 2,6 milliards d'euros les recettes de cette même branche en ne compensant ni la désocialisation des heures supplémentaires ni la baisse du forfait social ? Le Gouvernement a été prompt à à présenter ces mesures comme des cadeaux aux salariés et aux entreprises. Certains pourraient avoir le sentiment qu'on leur en présente désormais la facture Face à un État impécunieux et à un système de retraites en déséquilibre structurel, comment les différents régimes ayant accumulé des réserves pour garantir leurs engagements futurs pourraient-ils ne pas interpréter le régime universel comme une tentative de « hold-up »

et la confusion dans l'esprit de nos compatriotes lorsqu'il est question des retraites. Il a, hélas, parfaitement réussi, et ne doit donc pas s'étonner de récolter de la défiance eu égard aux promesses qu'il formule, en en termes de justice sociale et de maintien du pouvoir d'achat des retraités. Dans ce contexte, il est nécessaire que nous prenions le temps de faire le point sur le projet de réforme du Gouvernement, alors que s'achève la phase de concertation et que la rédaction de l'avant-projet de loi est presque finalisée. La formule de notre débat est vivante : après les interventions liminaires des représentants des différents groupes politiques, une séquence de questions-réponses s'engagera. nous permettre de balayer de nombreuses questions de nos concitoyens et des parlementaires que nous sommes. Reconnaissons-le, les sujets d'interrogation, voire d'inquiétude, ne manquent pas. Je pense aux conséquences du basculement du calcul des pensions en fonction des trimestres vers un système à points, singulièrement quand on a connu une carrière hachée en raison de périodes de chômage ou quand on s'est arrêté pour élever des enfants. Je pense à l'évolution du calcul des avantages familiaux, qui risque de pénaliser de nombreuses familles, tout particulièrement celles de trois enfants. Je pense à la transition pour les personnes relevant de l'un des régimes appelés à disparaître. Si l'on a beaucoup parlé d'un ou deux régimes spéciaux, bien davantage de personnes sont concernées, notamment les travailleurs indépendants. Je pense aussi à l'équilibre financier, car, à force de concessions discrètes et ciblées aux grévistes disposant des plus grandes capacités de nuisance, le Gouvernement pourrait bien réaliser l'exploit de proposer une réforme qui mécontente une majorité de Français, tout en plombant nos finances publiques.

Pourtant, au fil du temps, il s'est complexifié afin de s'organiser autour de logiques catégorielles. Ces logiques étaient respectables et cohérentes, car elles s'appliquaient à un temps où l'on cotisait à une même caisse toute sa vie. De ce système sont nés des régimes à différentes vitesses, créant des incompréhensions entre les Français. Et les réformes paramétriques, qui recherchaient presque toutes l'équilibre budgétaire, ont démultiplié la complexité et ont fini par opposer les Français au lieu de les unir. Oui, mes chers collègues, la défiance en notre système actuel de retraite est généralisée. Les seuls Français qui pensent sereinement à leur retraite sont ceux qui ont conservé le même travail toute leur vie et qui ont été inscrits à une caisse de retraite complémentaire avantageuse. Oui, je le répète, la défiance en notre système actuel de retraite est généralisée. Et pour cause ! Comment accepter de ne pas avoir les mêmes droits en fonction de la caisse à laquelle l'on cotise ? C'est ainsi que nous sapons la solidarité entre les générations, coeur du principe de répartition sur lequel repose notre système. Solidarité, simplification, équité, équilibre financier

Pour ce faire, cette réforme doit être systémique, tout en gardant son objectif d'équilibre financier à moyen terme. Citons quelques piliers qui en feront la stabilité l'universalité, avec un système unique de cotisations par points ; la solidarité, avec la suppression des 42 caisses et la volonté de conforter notre régime de répartition ; l'équité, car chaque euro travaillé donnera les mêmes droits à chacun une gouvernance ouverte qui garantira la prise en compte de tous, la stabilité à long terme et la certitude que la valeur du point et les pensions ne régresseront pas ; la protection des plus fragiles,

Le système universel fera cotiser chacun, à hauteur de 28 % de ses revenus, jusqu'à un plafond de 120 000 euros annuel, contre 324 000 euros actuellement. En d'autres termes, les droits à la retraite universelle par répartition s'établiront sur l'ensemble des revenus jusqu'à 120 000 euros par an. Au-delà, il sera demandé une cotisation de solidarité de 2,81 % qui ne donnera aucun droit à point de retraite, mais servira à la solidarité nationale. Les Français conçoivent que le système universel est le meilleur système, à la condition qu'il soit redistributif, solidaire et par répartition. Et c'est bien dans cette logique que les syndicats réformistes sont prêts à accompagner cette réforme. Pour autant, régime universel ne veut pas dire régime unique. Cela signifie qu'un euro cotisé, quel que soit le métier, ouvrira les mêmes droits. Parler d'universalité impose des réflexions sectorielles, et même des réflexions sur les spécificités de chacun, et demande des aménagements clairs et consensuels. C'est la raison pour laquelle un nouveau cycle de discussions s'est ouvert ce matin avec les organisations syndicales. se sont rassemblées aujourd'hui autour du Gouvernement pour lancer des travaux sur quatre objectifs qui font consensus, et qui sont centrés sur la pénibilité et les seniors. réunion, le Premier ministre a proposé aux partenaires sociaux un rendez-vous vendredi matin, afin de définir les contours de la conférence de financement de la future réforme des retraites, répondant ainsi positivement à la demande de Laurent Berger, secrétaire général de la CFDT. Ainsi, après plus de deux ans de concertations avec l'ensemble de nos concitoyens, en particulier avec les partenaires sociaux, il ne fait plus aucun doute que l'idée d'universalité, ainsi construite, est partagée. Alors, loin des débats politiciens- avec cette réforme, nous engageons tous les Français pour des dizaines et des dizaines d'années -, nous savons, en tant que sénateurs, que la cristallisation des mécontentements s'est opérée autour du seul volet paramétrique de cette réforme, l'âge d'équilibre à 64 ans. La proposition du Premier ministre est un premier pas, et notre débat peut apporter des éléments constructifs et consensuels permettant un compromis acceptable par toutes les parties. Mes chers collègues, je crois à la solidarité intergénérationnelle, je crois en notre système de répartition, je crois en la capacité de notre chambre de formuler des propositions positives qui seront à la hauteur de cette réforme que les Français méritent. La parole

mes chers collègues, à rendre hommage à tous ces salariés qui, depuis maintenant plus d'un mois, se mobilisent courageusement contre le projet de réforme des retraites, à travers un mouvement social de grande ampleur, largement soutenu par la population. d'État, votre gouvernement a décidé de faire passer en force cette réforme, sans concertation. Votre attitude est irresponsable

votre gouvernement a certes été contraint de descendre de sa tour d'ivoire ... Mais les pseudo-concessions accordées sont très loin de satisfaire la population. Au contraire, plus les membres de votre gouvernement y vont de leurs annonces, plus ils renforcent l'élan de solidarité interprofessionnelle, car plus personne n'est dupe. Tout le monde a bien compris en effet que cette réforme visait à obliger les salariés à travailler plus longtemps pour toucher moins de pension, d'autant que vous avez clairement annoncé votre volonté de bloquer les dépenses des retraites à 14 % du PIB. Avec des retraités plus nombreux et des dépenses bloquées, il faudra nous expliquer comment le montant des pensions ne baissera pas mécaniquement.

L'universalité, mise en avant, n'est qu'une illusion pour masquer le véritable objectif : niveler les droits sociaux vers le bas. Vous voulez d'abord inciter les salariés à travailler plus longtemps, avec un recul de l'âge de départ à la retraite à taux plein à 64 ans, voire au-delà, âge pivot ou pas. ou pas. Le Gouvernement va faire payer aux salariés son désengagement du financement des retraites. Les politiques successives que vous poursuivez- exonération de cotisations sociales et casse de l'emploi -entraînent un chômage de masse et minent les comptes de la sécurité sociale. Vous organisez le déficit de la sécurité sociale pour mieux la casser ! Vous vous attaquez également directement au montant des pensions de retraite. Vous le faites, d'une part, par le biais du système par points, un système bien connu des Suédois et des Allemands ; or les retraités de ces pays sont les plus pauvres d'Europe. Ce régime permet en effet d'ajuster la valeur du point en fonction des variations du marché. Ainsi, les salariés ne connaîtront le montant de leur pension qu'au moment de partir à la retraite, avec comme mauvaise surprise un faible revenu qui les incitera malheureusement à travailler plus pour augmenter Sincèrement, je pense que vous ne mesurez pas- ou alors vous n'en avez que faire -ce que cela représente, par exemple pour des ouvriers du bâtiment ou d'usine, des déménageurs ou des femmes de ménage, de travailler encore plus longtemps. d'autre part, en calculant le montant des pensions sur l'ensemble de la carrière des salariés du public comme du privé. Les salariés aux revenus modestes, dont la carrière a été entrecoupée de périodes de chômage, ceux qui sont entrés tard sur le marché du travail, ou encore les femmes, qui sont déjà pénalisées par les inégalités salariales et sociales, feront partie des plus grands perdants de votre réforme. Pour notre part, nous sommes dans le camp de ceux qui défendent le progrès social, et j'attire à ce titre votre attention sur la pétition concernant depuis dimanche, dont nous sommes signataires avec d'autres personnalités politiques et syndicales, de même que des artistes et des chercheurs. Nous vous demandons encore une fois de retirer votre projet de réforme de retraite par points et d'améliorer notre système de retraite par répartition sur ses bases actuelles. Nous avons des propositions, les syndicats vous ont aussi fait part des leurs, mais, évidemment, vous n'avez pas écouté ! En réponse, vous avez envoyé votre texte au Conseil d'État et l'avez inscrit à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale dès le 17 février. Véritable

Nous serons à leurs côtés dans la lutte pour exiger le retrait de votre projet de loi néfaste pour les salariés, toutes catégories confondues

le groupe Union Centriste, ainsi que l'ensemble des partis centristes, ont depuis longtemps milité pour une réforme universelle des retraites. Mais, il faut bien en convenir, si la préparation de cette réforme par Jean-Paul Delevoye fut exemplaire dans sa démarche- le Sénat y a d'ailleurs largement contribué

Rappelons tout d'abord qu'elle est nécessaire. Le système actuel est en perpétuelle recherche d'équilibre et génère trop d'inégalités. Il est injuste pour les personnes dont les carrières sont hachées, pour celles qui travaillent à temps partiel, pour les agriculteurs, pour les artisans et commerçants, pour les femmes, sans parler des pensions ainsi la proposition d'une retraite de base garantie à 1 000 euros par mois pour une carrière complète au SMIC. Rétablissons aussi la vérité pour tous ceux qui prétendent que le nouveau système sera par capitalisation. Une de plus ! Le système à points reste par répartition, c'est-à-dire que les actifs payent pour les pensions des retraités. Avec ce système, chaque heure travaillée donne des droits à la retraite, ce qui n'est pas le cas dans le mécanisme actuel.

tout d'abord que la valeur de service du point ne baissera pas. Elle sera indexée sur le salaire moyen, qui croît actuellement plus vite que le PIB. Les pensions continueront à augmenter au rythme de l'inflation, conformément à la loi de

Il n'y a pas plus bel exemple de réussite du paritarisme à la française. Faisons-lui confiance ! L'architecture du nouveau système, on le voit, est simple et claire. L'équilibre s'établit entre la valeur du point de cotisation, le nombre d'actifs, le montant des pensions et le nombre de retraités. Est-il besoin de faire des ajustements paramétriques

En clair, mettons pour l'instant entre parenthèses l'âge pivot. À ce propos, l'idée d'une conférence financière nationale évoquée par Laurent Berger rejoint la proposition avancée récemment par les présidents des groupes parlementaires centristes à l'Assemblée nationale et au Sénat.

quelques suggestions pour rassurer les salariés, en particulier ceux qui exercent des métiers pénibles. Les critères qui définissent la pénibilité sont précis, mais il faut les reconsidérer, notamment pour les charges lourdes.

toutefois une mise en garde : nous ne devons pas recréer de régimes spéciaux par branche ou entreprise. Les droits doivent être individuels ou par métier.

Une dernière recommandation concerne la transition entre les deux systèmes. Deux Français sur trois relèvent du secteur privé et un quart du secteur public, où il existe de fortes disparités entre professions

Ces propositions me paraissent de nature à redresser les contre-vérités, à calmer les inquiétudes légitimes, à rassurer le plus grand nombre et à sortir du conflit actuel. actuel. Il appartient maintenant au Parlement de graver dans le marbre de la loi ces principes et les nouvelles orientations pour un système universel plus équitable, plus juste et plus solidaire. Le Gouvernement serait bien inspiré, après avoir après avoir consulté et négocié avec les partenaires sociaux, d'écouter aussi le Parlement, notamment le Sénat, qui s'est beaucoup investi dans cette réforme. La parole est à M. La parole est à M. Patrick Kanner, pour le groupe socialiste et républicain.

Le Gouvernement, de son côté, se félicite d'une réforme des retraites bien calibrée, bien pensée, dont chaque point a été soupesé, disséqué, et qui a nécessité deux ans de travail En somme, la meilleure réforme qu'un gouvernement n'ait jamais portée ! Il n'y aurait pas d'impasse, pas de rejet et, de ce fait, pas d'inflexion non plus. C'est droit dans ses bottes de hussard que le Premier ministre mène ce travail, y compris en nous imposant une procédure accélérée. gouvernement, monsieur le secrétaire d'État, car, bien que représentants du prétendu nouveau monde, vous utilisez les mêmes vieilles recettes, les mêmes rengaines ! Rien de mieux pour décrédibiliser le mouvement social que dénoncer une minorité de privilégiés bloquant le pays pour conserver leurs avantages. Mais de quels privilégiés parle-t-on ? De ceux qui ne souhaitent pas partir toujours plus tard à la retraite, toujours moins dotés et en mauvaise santé ? Cela Cela m'ennuie de répéter devant vous, monsieur le secrétaire d'État, une chose que vous savez déjà, vous qui êtes un homme du Nord : un ouvrier a six ans d'espérance de vie de moins qu'un cadre. Quant à l'espérance de vie en bonne santé, c'est-à-dire sans incapacité, elle est de 64,5 ans pour les femmes et de 63,5 ans pour les hommes l'âge pivot à 64 ans est donc une aberration, une régression sociale ! Mais ce n'est pas la seule ligne rouge pour nous. Avec la réforme qui se profile, l'ouvrier qui a les conditions de travail les plus pénibles ne partira pas plus tôt à la retraite que le cadre. Il ne récupérera jamais les six ans d'écart d'espérance de vie. Les plus modestes paieront la retraite des plus favorisés. Et on nous parle d'égalité cette réforme est structurellement inégalitaire. Et pour viser l'égalité et la justice sociale, il ne suffira pas de moduler l'âge pivot ni même de reculer sur ce paramètre financier. Il faut revoir la prise en compte de la pénibilité. Rappelons à cet égard qu'une des premières mesures d'Emmanuel Macron a consisté à revenir sur les dix critères de pénibilité mis en oeuvre sous le précédent quinquennat au profit des salariés que le travail use. Le Medef- le Medef ! -les trouvait trop compliqués- traduction : trop favorables aux salariés ... Le Gouvernement a réduit ces critères à six. Désormais, pour pouvoir bénéficier d'un départ à la retraite quand on est exposé aux facteurs de pénibilité, il faut soit être victime d'invalidité soit souffrir d'une maladie professionnelle, donc avoir dit définitivement adieu à une retraite en bonne santé. Car à quoi servaient ces dix critères du compte pénibilité ? À acquérir des droits spécifiques à la formation pour évoluer professionnellement, à réduire son temps de travail en fin de carrière ou sa durée d'activité pour partir plus tôt à la retraite.

c'est parce que nous avons pris nos responsabilités et réussi à sauver notre système universel de retraite par répartition avec la réforme Touraine que nous pouvons dire aujourd'hui qu'une autre voie est possible. Le système actuel est naturellement perfectible. Il peut et doit encore évoluer, mais l'argument d'autorité employé par le Gouvernement est un leurre. Il n'y a pas d'urgence à réformer du fait d'un prétendu sous-financement du système des retraites, et encore moins de le faire dans ces termes.

prise en compte de la pénibilité et des carrières longues qui doivent être au centre d'une réforme de justice ; amélioration de l'égalité entre les hommes et les femmes, en renforçant prioritairement l'acquisition de droits à la retraite pour les carrières discontinues et les droits dérivés. Parce que niveau de vie et espérance de vie sont fortement corrélés, le financement du système de retraite doit responsabiliser davantage les entreprises en fonction de leur politique en matière de pénibilité et de santé au travail, ainsi que les salariés percevant de hauts revenus puisqu'ils sont le plus longtemps à la retraite. Ces nouvelles sources de financement doivent permettre de garantir à moyen et long terme le niveau de vie des retraités. Tels sont les axes de progrès social que nous entendons soumettre au débat. Entendez-nous, monsieur le secrétaire d'État ! Ne méprisez pas les Français, ne méprisez pas le Parlement ! Votre réforme devait rassurer : c'est déjà un échec de ce point de vue. Le climat de régression sociale dans lequel vous menez vos travaux ne peut qu'accentuer la déchirure du tissu social. Réformer le système de retraite, c'est refonder le pacte social. Quand allez-vous écouter la population pour présenter un projet d'avenir, un projet de confiance, un projet de justice sociale ? Votre projet à l'impact indéterminé, systématiquement et paramétriquement incontrôlé, est fondamentalement injuste. Monsieur le secrétaire d'État,

Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, en 1945, le Conseil national de la Résistance souhaitait déjà donner une retraite permettant aux vieux travailleurs de finir dignement leurs jours. Bien plus qu'un acquis social, notre système de retraite par répartition incarne les valeurs humanistes chères au groupe RDSE et qui sont au coeur du pacte républicain. Soixante-quinze ans plus tard, ce pilier de notre équilibre social est de plus en plus fragilisé par une évolution démographique défavorable et un déficit qui pourrait devenir important. Selon les prévisions du COR, le régime serait déficitaire de 8 à 17 milliards d'euros en 2025 et la trajectoire se dégraderait jusqu'en 2030. Cette situation ne date malheureusement pas d'hier. En préface du Livre blanc sur les retraites, Michel Rocard rappelait : « Nous avons [ ...] vis-à-vis des générations futures un devoir de lucidité et un impératif de solidarité. Nous leur devons des choix pour garantir leur avenir. » C'était en 1991 Cela fait bientôt trente ans que les gouvernements successifs, de gauche comme de droite, tentent d'apporter des réponses satisfaisantes- en vain ! Et cela fait plusieurs années que nos concitoyens, notamment les jeunes, sont particulièrement inquiets quant à l'avenir du système actuel. Ce dossier est en instance depuis trop longtemps. Oui, une réforme de notre système de retraite est évidemment nécessaire. En effet, ne rien faire menacerait la pérennité de notre régime par répartition et hypothéquerait l'avenir des générations futures. On ne peut se permettre de faire peser sur ces générations tout le poids du financement de nos retraites ; cela ne serait pas raisonnable. Comme l'a récemment rappelé le président Jean-Claude Requier dans cet hémicycle, ne rien faire serait tout simplement irresponsable. Nos concitoyens ne comprendraient pas que nous n'ayons trouvé ni le temps ni les mots d'une réforme juste. C'est pourquoi nous notons la volonté du Gouvernement

Toutefois, comme nous le rappellent nos concitoyens dans le cadre des grèves qui durent depuis plus d'un mois, la méthode du Gouvernement pose question et nous avons surtout besoin de plus de clarté sur le financement des futures retraites. Cette réforme ne doit pas être synonyme de rupture sociale ni de paupérisation des Français. Oui, monsieur le secrétaire d'État, une réforme systémique est nécessaire et le souhait du Gouvernement de mettre en place un système qui repose sur trois grands principes- l'universalité, l'équité et la responsabilité -est honorable. Ainsi, pour garantir la pérennité et l'universalité de notre système de retraite, il est souhaitable d'adopter un régime identique dans ses fondements pour tous les Français. C'est sans doute l'utilisation du terme « universel » qui crée autant d'incompréhension dans la population. Cependant, un système équitable doit permettre de mieux protéger nos concitoyens, en tenant compte notamment des périodes de maternité, des carrières heurtées ou de la pénibilité qui, pour nous, est un élément essentiel qu'il faut prendre À titre d'exemple, comment imaginer qu'un marin pêcheur doive travailler jusqu'à 64 ans, comme le suggère dans son état actuel le projet du Gouvernement ? Dès lors, comment peut-on raisonnablement penser qu'un euro puisse ouvrir les mêmes droits pour tous ? Par ailleurs, le pacte originel imaginé en 1945 par le Conseil national de la Résistance prévoyait le maintien des régimes spéciaux antérieurs pour une période provisoire. Le COR s'est lui-même interrogé à plusieurs reprises sur la simplification de notre système de retraite particulièrement complexe. Ainsi, votre projet d'alignement des régimes spéciaux semble s'inscrire dans cette logique historique. Mais est-ce pour autant possible ? Cette réforme suscite une réelle inquiétude, la défiance, le mécontentement et la colère d'une partie de nos concitoyens. Aussi, pour sortir de l'impasse, plusieurs secteurs ont obtenu des aménagements, voire le maintien de leur spécificité. Les régimes spéciaux laisseraient ainsi la place à des régimes « spécifiques », mais basés sur quelle universalité ? Lors d'un débat sur la réforme des retraites à Rodez le 3 octobre dernier, le Président de la République avait affirmé qu'il n'accepterait aucune exception dans son futur régime universel de retraite. Et lors de ses voeux aux Français, le 31 décembre, il a de nouveau rappelé que ce projet était un projet de justice et de progrès social, parce qu'il assurait l'universalité.

Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, Bismarck disait : « Les lois, c'est comme les saucisses, il vaut mieux ne pas savoir comment elles sont préparées. » Mais les Français ne sont pas comme Bismarck, ils préfèrent le savoir. Et nous, parlementaires, encore plus. D'où l'utilité de ce débat, monsieur le président de la commission des affaires sociales. Lorsqu'un gouvernement décide une réforme des retraites, monsieur le secrétaire d'État, on sait d'avance qu'il y aura des bosses sur la route. En France, la réforme porte en elle la grève comme la nuée l'orage. Notre pays est donc reparti pour une nouvelle crise de nerfs, énième tentative de de 1789 qui menace désormais de se renouveler tous les ans. Vous avez les grèves et les manifs, comme Juppé en 1995, Raffarin en 2003, Villepin en 2006, Fillon en 2010, El Khomri en 2016, Macron l'an dernier- enfin un sport où nous sommes champions du monde incontestés ... Marx disait que l'histoire se répète, la première fois comme une tragédie, la deuxième comme une farce ; mais au vingt-cinquième épisode, ce n'est plus une farce, c'est une série Netflix- en l'occurrence une mauvaise ... Les grèves, c'est long, surtout vers la fin, et surtout pour ceux qui les subissent, mais les bloqueurs se moquent de ceux qui les subissent. Et voilà comment le pays est aujourd'hui en marche, mais en marche arrière, et comment depuis un mois les Français sont en marche, mais à pied Au moment où, dans le calme, nos voisins européens ont tiré les conséquences de l'allongement de la vie en instaurant la retraite à 65 ans, en France, les démagogues du Rassemblement antinational, de la France soumise à Cuba et de la CGT proposent la retraite à 60 ans. Pour eux, l'argent public, c'est comme l'eau bénite, tout le monde se sert. Mais à part eux, tous les Français savent que la réforme est inéluctable : déséquilibre démographique, déficit structurel, inégalités criantes sont des épées de Damoclès qui pèsent sur les retraités et sur les futurs retraités dans un pays où le système coûte 14 % du PIB contre 10 % en moyenne en Europe. une majorité de nos concitoyens est plutôt favorable à l'universalité du nouveau système, aux mesures en faveur des femmes, des agriculteurs, des titulaires de petites retraites ou de ceux qui ont une carrière hachée et à la suppression des régimes spéciaux pour lesquels les Français qui partent à la retraite en moyenne à 63,5 ans payent 8 milliards d'euros afin que d'autres y partent à 52 ou 57 ans. Alors, pourquoi une telle confusion aujourd'hui ? Pas seulement parce que nous sommes, dit-on, des « Gaulois réfractaires » ni même parce que la CGT a pour devise « Je bloque, donc je suis », mais aussi parce que le service après-vente a connu des ratés. Le Gouvernement a réussi à rassembler, mais hélas contre lui, en suivant une ligne droite qui a beaucoup zigzagué. Je ne lui jette pas la pierre puisque, comme je le disais, chaque réforme depuis cinquante ans met des centaines de milliers de gens dans la rue et personne n'a jamais trouvé la recette pour l'éviter. Nous aimerions donc quelques clarifications. Notre première inquiétude, c'est de voir chaque étape de la négociation augmenter la facture. Nous voudrions connaître le chiffrage exact de la hausse des dépenses publiques induite par toutes les mesures nouvelles annoncées chaque jour. Bien sûr, le Premier ministre a raison de refuser la distinction purement fictive entre réformes systémique et paramétrique ; le système doit être équilibré sur le long terme comme sur le court terme- c'est une évidence. Âge pivot ou augmentation pure et simple de l'âge de départ, c'est un débat assez académique à mes yeux. Je crains seulement que dire qu'on va faire cette réforme en l'équilibrant grâce au seul âge pivot, et sans lui, ce soit comme prétendre qu'on va faire rentrer un édredon dans une valise. Il va falloir nous expliquer comment. Deuxième inquiétude, les concessions qui s'accumulent à chaque rencontre avec les partenaires sociaux et qui ont abouti dans les faits au maintien de plusieurs régimes particuliers, souvent justifiés, sont-elles terminées ? Ou bien va-t-on, à travers les mesures de compensation demandées à la RATP et à la SNCF, les faire payer par des entreprises qui cumulent la sous-rentabilité, le surendettement, l'effondrement de la qualité des services rendus et le sous-investissement ?

Si ces réserves, fruits de l'épargne et d'une bonne gestion, devaient devenir la variable d'ajustement d'une facture trop lourde, j'ai peur que de nombreuses personnes qui vous sont plutôt favorables ne deviennent quelque peu courroucées. Monsieur le secrétaire d'État, cette réforme est indispensable et il faut savoir gré au Gouvernement de l'avoir lancée. Nous souhaitons pouvoir la voter, comme le Sénat l'a fait pour d'autres depuis deux ans- le code du travail, l'école ou le statut des cheminots -, mais notre grande question à ce stade, c'est : quelle réforme exactement ? Vous l'avez compris, nous voulons savoir comment sont fabriquées les saucisses, mais nous souhaitons aussi qu'à la sortie elles ne soient pas saucissonnées.

nombreux rapports, préconisations, débats et colloques. Au fil des réformes précédentes, les gouvernements successifs et les partenaires sociaux ont dû prendre des décisions importantes, parfois difficiles,

et au-delà, de nombreux pays ont ouvert le débat sur la protection sociale. Il en ressort deux modèles radicalement distincts : l'individualisation et l'assurance, d'une part, le collectif et la mutualisation, d'autre part. C'est résolument ce second choix que le Gouvernement a fait et, conformément à l'engagement que le Président de la République a pris devant les Français et les Françaises en 2017, c'est dans ce sens que nous voulons construire la grande transformation de notre système de retraite.

par leurs cotisations les retraites d'aujourd'hui. Pour y parvenir et parce que nous avons mis le dialogue social au centre de notre action, les travaux menés par Jean-Paul Delevoye

elles ont conforté la conviction du Gouvernement de rassembler les Français autour de trois principes qui constituent le coeur du système universel de retraite. : l'universalité. Elle garantira une protection sociale plus forte et plus durable, parce qu'elle ne dépendra plus de la démographie de chaque profession. Elle assurera aussi une plus grande liberté et une meilleure mobilité professionnelle.

l'équité et la justice sociale pour faire en sorte de marquer une solidarité forte de notre pays vis-à-vis des Français les plus fragiles. Le président Kanner s'en inquiétait tout à l'heure- il parlait d'une « trappe à pauvreté » -, mais il doit savoir que le projet du Gouvernement prévoit une pension minimale d'au moins 85 % du SMIC net pour une carrière complète

responsabilité d'être lucide sur notre évolution démographique. Fidèle à l'engagement du Président de la République, le Gouvernement ne reviendra pas sur l'âge légal de départ à la retraite qui sera maintenu à 62 ans, mais il fait aussi le choix de la liberté individuelle, en incitant les Français à travailler un peu plus longtemps dans le but de garantir les pensions et de financer un niveau élevé de solidarité.

Pour toutes les générations, nous gardons le même principe de justice : les règles changeront pour les citoyens qui sont en 2020 à plus de dix-sept ans du départ à la retraite.

Nous allons procéder au débat sous la forme d'une série de questions-réponses dont les modalités ont été fixées par la conférence des présidents.

J'en veux pour preuve le principe du calcul par points pour les droits à la retraite réclamé par la CFDT. Quant au syndicalisme de politiques, il joue de la posture nationale sans être investi par le suffrage universel et sombre dans l'excès J'en veux pour preuve des syndicats qui s'opposent, par principe, à la réforme et refusent toute négociation, allant jusqu'à utiliser des moyens de pression illégaux, comme le blocage de raffineries, les coupures d'électricité, ou des menaces sur des collègues voulant travailler. On va pleurer ! Il n'y a rien de durable qui se construise dans l'excès ! Au-delà du débat sur la retraite universelle, l'avenir du syndicalisme se joue et nous devons le préserver ! Ne sombrons pas dans l'exemple britannique qui, à force de promouvoir un syndicalisme de politiques, a précipité sa chute. Aujourd'hui, le point d'achoppement se trouve dans la réflexion sur l'équilibre financier du système de retraite. Laurent Berger, au nom de la CFDT, a proposé la tenue d'une conférence de financement. En agissant ainsi, il défend les intérêts des salariés et respecte notre démocratie. Montrer que le Gouvernement peut travailler avec lui doit constituer un signal fort, non seulement pour mener à bien cette réforme, mais aussi pour préserver l'avenir du syndicalisme. C'est dans ce champ qu'il faut se situer, et non dans celui du politique. J'invite ceux qui se placent dans cette posture à se soumettre au suffrage universel et, ensuite, à proposer des lois.

Cette vision passéiste est contredite par les progrès de la médecine, par ceux de la recherche, par les bouleversements dans la société et les rapports sociaux. Ceux-ci portent en eux de nouveaux progrès pour l'humanité, pour peu qu'ils soient mis au service de la justice, du bien commun, et non du profit au bénéfice de quelques-uns. Ainsi, la retraite est vécue non plus comme la fin de la vie, mais comme le début d'une nouvelle vie, hors travail, riche d'activités et de découvertes. Ce n'est pas une charge ; c'est un progrès pour la société, un projet de civilisation

Voici quelques exemples de propositions. Mettre fin au régime spécial des revenus du capital, qui ne participent pas ou participent insuffisamment au financement des retraites, en alignant le taux de cotisation sur celui des revenus du travail, rapporterait 31 milliards d'euros.

Monsieur le secrétaire d'État, allez-vous enfin retirer cette réforme massivement rejetée et accepter de débattre des alternatives et des financements qui les accompagnent ?

au sein du monde rural. Des revendications soutenues de longue date par les agriculteurs devraient figurer dans le texte définitif, notamment un système par points minimale à 85 % du SMIC pour une carrière pleine. De même, les avancées concernant le cumul entre activité et retraite, ainsi que la fin des conditions de ressources pour la pension de réversion sont autant de bonnes nouvelles pour la profession. ces mesures, dont nous espérons qu'elles seront effectivement retenues dans la version présentée en conseil des ministres à la fin du mois, ne concernent pas la majorité des agriculteurs déjà à la retraite

terme, de retrouver la confiance. Mais il ne faut pas oublier de répondre à la situation d'urgence, parfois de détresse, dans laquelle se trouvent de nombreux agriculteurs, artisans et personnes ayant connu des carrières hachées. La

En vertu du principe de solidarité nationale, l'État verse chaque année 6,2 milliards d'euros à dix régimes spéciaux déficitaires, qui sont principalement ceux de la SNCF, de la RATP, des marins et des mines. Ces régimes spéciaux sont déficitaires en raison de leur déséquilibre démographique : il n'y a plus assez d'actifs, donc de cotisations, pour couvrir les pensions des retraités. Il est par conséquent nécessaire et légitime que l'État comble le manque de contributions.

qui les financeront. Pas la collectivité ». J'en viens donc aux deux régimes spéciaux de la SNCF et de la RATP, pour lesquels la contribution de l'État s'élève à plus de 4 milliards d'euros. Dans un récent rapport, la Cour des comptes a estimé que, sur ce total de 4 milliards d'euros, l'État finançait 300 millions d'euros d'avantages spécifiques à la RATP et 600 millions d'euros à la SNCF. Ce montant annuel de 900 millions d'euros n'a rien à voir avec la légitime compensation démographique. Il finance des avantages spécifiques propres à ces deux régimes. Monsieur le secrétaire d'État, est-ce à la solidarité nationale d'honorer ces sommes ? En cohérence avec vos propos concernant les pilotes de ligne, à travers lesquels vous affirmez que l'État ne paiera pas les suppléments au régime universel, allez-vous retirer à la SNCF et à la RATP ces 900 millions d'euros d'avantages spécifiques ?

! Malgré cela, nous venons de passer quasiment six mois sans que le Gouvernement soit capable de préciser quels sont les enjeux budgétaires. C'est pourtant là la question principale

Donnez-moi un ordre de grandeur ! Je vous demande non pas de m'expliquer comment vous allez régler le problème- vous allez me répondre que les négociations sont en cours avec les partenaires sociaux -, mais simplement de me donner un ordre de grandeur

ces propos sont ceux du Président de la République lors de l'audience solennelle de la rentrée de la Cour des comptes le 22 janvier 2018. D'où vient, dès lors, cet acharnement à vouloir imposer un âge pivot ? Après les annonces du Premier ministre sur la future réforme, les services ont sorti des pseudo-simulateurs, censés donner des indications aux citoyens sur leurs droits futurs. En fait, il s'agirait plutôt de pratiques divinatoires, tant il est aléatoire de prévoir une situation pour des gens qui ont aujourd'hui la vingtaine

il travaille depuis l'âge de 19 ans. Grâce aux services en ligne de sa caisse de retraite, il sait qu'il pourra faire valoir ses droits à la retraite à 62 ans, car il aura alors atteint l'âge légal de départ et comptera le nombre de trimestres requis. Il sait aussi qu'il percevra une retraite d'un montant de 1 400 euros. Que se passera-t-il pour lui si un âge d'équilibre à 64 ans est mis en place entre-temps ? Première solution, Jean travaille deux ans de plus pour conserver une retraite à taux plein, sachant qu'il travaille déjà depuis 43 ans. solution, Jean décide de faire valoir ses droits à 62 ans et perdrait jusqu'à 140 euros mensuels, et ce définitivement. À ce niveau de revenu, 140 euros en moins, ça fait réfléchir Pile, Jean perd ; face, il ne gagne pas ! C'est, monsieur le secrétaire d'État, le seul simulateur crédible aujourd'hui ! Jean fera partie de cette cohorte de salariés qui auront largement contribué au financement des retraites et à qui on demandera de contribuer encore et encore Mais tout cela va se discuter, n'est-ce pas, monsieur le secrétaire d'État ? C'est ce que le Gouvernement clame Ça va tellement se discuter que vous fermez systématiquement la porte à toutes les demandes syndicales de retrait de l'âge pivot

d'ailleurs, que nous assistons cette semaine enfin à une véritable discussion entre le Gouvernement et les partenaires sociaux, et ce depuis l'engagement du conflit. Pourtant, depuis deux ans, les choses semblaient bien engagées ... tout au moins en apparence

Malgré cette perspective louable, aucune réponse satisfaisante n'est apportée à cette question dans les débats actuels sur la réforme. J'irai même plus loin en disant que tout élu responsable doit, en abordant une réforme quelle qu'elle soit, s'assurer d'abord des modalités de son financement et des conséquences qu'elles peuvent entraîner. À cet égard, j'ai pu noter que le Gouvernement allait mettre en ligne un simulateur, qui permettra aux Français, en théorie, de mesurer l'impact personnel de la réforme, telle qu'elle est envisagée. Pourtant, dans le flou régnant en l'espèce, cela risque d'être la quadrature du cercle. Mais ce n'est pas le sujet de ma question ... Ce mardi, le Gouvernement s'est dit prêt à envisager la tenue d'une conférence de financement de la réforme, comme le suggère la CFDT, dissociant de fait la réforme de son financement.

qui siègent dans cet hémicycle sont des élus responsables. Pour preuve, je vous renvoie tout simplement à ce qui s'est passé lors de l'examen du PLFSS, notamment à propos du plan Hôpital : nous avons refusé de statuer alors que des discussions étaient en cours. Pensez-vous réellement que nous allons travailler sur un projet de texte

En tout premier lieu, je veux une nouvelle fois évoquer l'absence de politique familiale qui, de mon point de vue, est une politique d'investissement dans l'avenir face au vieillissement de la population. Avouons-le, aujourd'hui, rien n'encourage et n'accompagne les jeunes couples à devenir parents. Or sans futurs cotisants, il sera plus difficile de maintenir une solidarité intergénérationnelle au moment de la retraite. C'est pourquoi il conviendrait de s'interroger sur la baisse de 8,5 % en dix ans du nombre de naissances. Par ailleurs, le Premier ministre assure que les femmes seront « les grandes gagnantes de la réforme ». Laissez-moi avoir quelques doutes, car elles seront les grandes gagnantes si elles restent en couple. Or près d'un mariage sur deux se conclut par un divorce. Les femmes touchent en moyenne un salaire inférieur de 26 % à celui des hommes, et c'est encore pire pour ce qui concerne leur pension de retraite, puisque celle-ci est inférieure de 42 % à celle des hommes. En raison de ces inégalités salariales, les familles appliqueront la majoration de 5 % de la pension perçue dès le premier enfant au salaire des hommes, bien sûr. À partir du moment où l'homme gagne davantage, il est plus judicieux, d'un point

est d'autant plus regrettable avec la réforme en prévision des pensions de réversion. Si la future réforme sera plus avantageuse en garantissant au conjoint survivant 70 % des ressources du couple, cette garantie est soumise à une condition : que le couple soit marié. Cette condition exclura donc les couples divorcés, alors qu'aujourd'hui la pension de réversion et partagée au prorata de la durée du mariage. Monsieur le secrétaire d'État, comment comptez-vous résorber l'écart de pension que pourront subir les femmes avec cette réforme ? Quelle place donnez-vous à la politique familiale dans cette dernière ?

Premièrement, aujourd'hui, les pensions de réversion sont versées dès 55 ans aux veufs et aux veuves, lesquelles sont le plus souvent concernées. Confirmez-vous que, selon votre projet, les veuves devraient désormais attendre 64 ans, soit neuf ans de plus, pour toucher leur pension de réversion ? Deuxièmement, trouvez-vous juste d'exclure les ex-conjoints divorcés du bénéfice de la pension de réversion ? Il n'est pas rare que des femmes qui ont vécu pendant vingt-cinq ans avec un homme et n'ont pas ou peu travaillé pour élever leurs enfants soient amenées à divorcer tardivement. Ne craignez-vous pas que l'exclusion des femmes divorcées du bénéfice de la pension de réversion n'accroisse la dépendance économique des femmes à l'égard de leur mari, particulièrement en cas de violences conjugales ? Troisièmement, vous mettez en avant votre volonté de relever à 1 000 euros le montant minimal de pension, mais, si j'ai bien compris, à condition que la carrière ait été complète. Pour ma part, je n'ai toujours pas compris ce qu'est une carrière complète dans un système à points. Pouvez-vous nous le dire

réduire les pensions des femmes fonctionnaires et, dans le même temps, prétendre que votre réforme ne va pas pénaliser les femmes

Vous n'avez pas répondu pour ce qui concerne l'exclusion des femmes divorcées des pensions de réversion. Or vous exposez les femmes aux violences conjugales en les maintenant dans la dépendance économique de leur mari. Vous n'avez pas non plus répondu à propos des femmes fonctionnaires. En fait, vous n'avez répondu à aucune des quatre questions que je vous ai posées. M. René-Paul Savary, pour le groupe Les Républicains.

Monsieur le secrétaire d'État, c'est à tort que vous invoquez la justice sociale pour justifier votre réforme des retraites. Notre système actuel unique ne nécessitait que des aménagements pour devenir encore plus juste, voire universel. C'est à tort que vous revendiquez l'esprit du CNR, qui aspirait, après les horreurs, à une société plus harmonieuse, plus épanouissante. Votre réforme, au contraire, détricote le collectif, et votre projet n'a plus de répartition que le nom. Chacun paie pour lui. Les conséquences de votre réforme seraient terribles. J'ai pris le temps d'effectuer une simulation comparative à partir de chiffres que vous ne contesterez pas, car ce sont les vôtres- sauf erreur -, sortis de votre simulateur. J'ai conjugué deux de vos exemples avec des carrières linéaires sans interruption, sans bas salaires, sans galères pour le premier emploi, sans période de chômage ni de maternité ; bref, le paradis

moins 1 000 euros par mois. Comme les carrières linéaires n'existeront plus, comme le premier emploi sera difficile à trouver, ceux qui commenceront à un niveau bas, qui auront des carrières hachées, soit la quasi-totalité de la population, auront commis le péché originel qu'ils devront payer jusqu'à la fin de leur vie. C'est la condamnation des efforts de de qualification et de formation

car la question des retraites est non pas une question technique, mais une question sociale importante, qui correspond à l'effort de toute une vie de travail et qui touche à l'avenir de nos aînés. Sur ce sujet majeur, les Français ont le droit à un débat clair et honnête ; vous leur devez. Le Premier ministre a mis en avant un certain nombre de mesures qui étaient attendues, notamment par ceux qui travaillent dur et gagnent peu. Je pense au minimum contributif des salariés du privé et des régimes alignés, qui serait porté à 1 000 euros en 2022. Ce complément de pension serait attribué aux assurés qui ont travaillé durant leur vie active, afin qu'ils gagnent un peu mieux que le minimum vieillesse accordé aux personnes qui n'ont pas cotisé. Cette retraite à 1 000 euros est indispensable eu égard à la justice, l'équité et la solidarité envers nos aînés, dont certains se retrouvent sous le seuil de pauvreté. Qui aujourd'hui peut trouver normal de percevoir une faible pension après une vie de travail ? La question du travail est d'ailleurs essentielle dans ce débat sur les retraites : pour pérenniser notre système de retraite par répartition, il faut promouvoir le travail tout au long de la vie pour garantir un équilibre entre actifs et cotisants. Nous devons revaloriser du travail dans la société. Cela passe aussi par la revalorisation des pensions de retraite. Alors que les droits sont nettement plus faibles dans certains régimes, comme ceux des artisans, des commerçants et des professionnels du monde agricole- la majorité d'entre eux touchent de faibles pensions, notamment en raison de carrières incomplètes -, il ne faudrait pas que la retraite à 1 000 euros devienne un leurre, d'autant qu'elle a été très longtemps repoussée. Monsieur le secrétaire d'État, pouvez-vous nous confirmer que cette mesure s'appliquera réellement ? Quelles en seront les modalités ? Quelles seront les interférences avec les retraites complémentaires ? La parole est à M.

poser. Elle risque de paraître minime par rapport aux grandes inquiétudes et aux questionnements qui ont été évoqués depuis le début de ce débat. En effet, en tant que président du groupe d'études sur les pratiques sportives et les grands événements sportifs, je souhaite aborder la question

des revenus qui avoisinent les 1 000 euros par mois. Le PLFSS pour 2012 a introduit dans la loi un dispositif spécifique d'ouverture de droit à la retraite pour les sportifs de haut niveau. Relevant du régime général de la sécurité sociale, sous certaines conditions de ressources et d'âge, bénéficient de la validation de trimestres- jusqu'à seize trimestres, soit une olympiade -correspondant à un revenu fictif d'environ 1 500 euros par mois. Par ailleurs, ce même PLFSS prévoyait qu'avant le 1 octobre 2013 le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant le coût du dispositif prévu et étudiant la possibilité d'augmenter le nombre de trimestres. Comme souvent, ce rapport n'a pas été rendu ... Monsieur le secrétaire d'État, comment comptez-vous traiter le cas de ces sportifs de haut niveau dans le cadre de la réforme des retraites qui sera prochainement examinée ?

le désordre organisé, des saccages perpétrés et 12 milliards d'euros dépensés pour acheter la paix sociale, voilà maintenant la vie en rouge ! Le chaudron est de nouveau en ébullition, et j'évoque malheureusement non pas le stade Geoffroy-Guichard, cher à notre collègue Bernard Bonne, mais notre beau pays et sa réforme des retraites Que nous disaient le candidat Emmanuel Macron et sa majorité en 2017 ? « Notre projet est de clarifier et de stabiliser les règles du jeu une fois pour toutes en mettant en place un système universel, juste, transparent et fiable, dans lequel chacun bénéficie des mêmes droits. Qui peut raisonnablement être contre un tel objectif ? En revanche, s'agissant de la méthode, vous repasserez ! Après avoir satellisé pendant dix mois M. Delevoye, votre prédécesseur, dont on se demande encore avec qui il a dialogué en France pendant tout ce temps pour aboutir à une telle impasse, après les conclusions dithyrambiques du désormais fameux Conseil d'orientation des retraites selon lequel « les perspectives financières permettent d'envisager l'avenir avec une sérénité raisonnable »- à la bonne heure !

Les partenaires sociaux des deux régimes de retraite complémentaires du secteur privé Agirc-Arrco, fusionnés en 2019, ont été capables, eux, de signer, le 30 octobre 2015, un accord national permettant d'envisager un retour à l'équilibre des comptes pour 2020. Quand allez-vous vous résoudre à adopter une méthode semblable et crédible, afin que ce triste épisode cesse dans notre pays et que nous retrouvions enfin la vie en rose à laquelle nous aspirons tous ?

d'une séance de questions tout à fait intéressante, même si nous n'avons pas toujours obtenu de réponses, ce que nous pouvons tout à fait comprendre. Sachez que nous continuons à travailler et que, quelles que soient nos différences, nous arrivons à faire des propositions